Mes chers collègues, les conclusions adoptées par la conférence des présidents, réunie ce jour sont consultables sur le site du Sénat, elles seront considérées comme adopté en l'absence d'observation, d'ici la fin de la séance, l'ordre du jour appelle en application de l'article 16 bis alinéa 2 du règlement, la proposition de création d'une commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique, sous réserve de sa transmission je soumets donc cette proposition au Sénat, il n'y a pas d'opposition. Il en est ainsi décidé. Conformément à la décision de la conférence des présidents, la désignation des 37 membres de cette commission spéciale aura lieu en séance publique, demain à 16 nous reprenons la discussion du projet de loi relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique dans la discussion des articles, nous sommes parvenus à l'amendement numéro 247 rectifié tendant pas insérer

présenté par Monsieur Gold de monsieur Gold. Merci madame la présidente, monsieur le ministre, chers collègues, cet amendement de notre collègue Bertrand a pour objet de mieux représenter les communes déléguées au sein des communes nouvelles au sein des communes nouvelles la représentativité à long terme des communes déléguées n'est pas assurée en effet dans une commune nouvelle de plus de 1000 habitants où le mode de scrutin pour les élections municipales est un scrutin de liste, rien n'oblige les candidats têtes de liste à prendre des représentants de toutes les communes déléguées en position éligible, ce voeu de représentativité des communes déléguées au sein des communes nouvelles et souvent exprimée dans les chartes des communes nouvelles mais sans avoir un quelconque caractère obligatoire, or la représentativité des communes déléguées au sein des communes nouvelles est un point de blocage pour beaucoup de petites communes dans leurs démarches visant à la création d'une commune nouvelle cette proposition de loi tendant à garantir la représentation des communes déléguées au sein des communes nouvelles introduirait plusieurs changements dans les communes nouvelles de plus de 1000 habitants, la liste des candidats devrait être composée de candidats résidant dans chaque commune, déléguée le maire délégué devrait être choisi parmi les conseillers municipaux résidant dans la commune, déléguée et enfin un conseiller municipal ne pourraient être remplacés que par un candidat résidant dans la même commune déléguée que lui, je vous remercie. Merci monsieur Gold madame la rapporteure, avis de la commission. d'une liste de candidats aux municipales dans les communes nouvelles où il existe des communes déléguées donc vous proposer que la loi organise la représentation de chacune des communes déléguées pour veiller à ce que l'ensemble des territoires soit bien représentés, on a déjà eu l'occasion avec notre collègue Bertrand d'évoquer les sujets au travers d'une PPL qui l'avait déposée. Je comprends tout à fait l'acquisition et que je n'imagine pas qu'un candidat à des municipales au titre du une nouvelle écarte de de ces 2 listes des communes déléguées et votre proposition pose à enfin peut poser un problème, imaginons une commune nouvelle faite de 2 communes ont décidé de la loi organise la représentation de chacune des communes, vous avez un candidat qui, au moment des élections municipales se présentent au titre de la commune, ah, ah, parce qu'il y réside donc il sera considéré comme appartenant au quota des candidats de la commune à à 6 mois après il déménage, il va habiter dans la commune B mais toujours au sein de la commune nouvelle comment considère-t-on les choses est-ce que ça veut dire qu'il perd son siège puisqu'il en a été élu au titre de la commune à dont il aurait déménagé, on est dans une impossibilité réelle d'organiser les choses, toutefois, la commune nouvelle qui est un projet, on va dire de nouvelles communes doit. S'organiser d'une manière un peu par paliers pour réussir un vrai projet de territoire et je pense que les chartes qui existe aujourd'hui, alors vous avez raison, elles n'ont pas une valeur légale, mais elles font partie du consensus, d'un projet de territoire et je crois qu'elles engagent chacun des des conseillers municipaux et tout particulièrement les mères et moi je suis assez confiante pour que sur la plupart des communes nouvelles, les choses s'organisent une manière favorable ancrer ces difficultés, donc c'est une demande de retrait ou un avis défavorable. Merci madame la rapporteure, monsieur le ministre. Oui, madame la présidente, même avis que la commission.

2 amendements qui font l'objet d'une discussion commune le 1er le 907 rectifié bis Monsieur Jacquin, vous avez la parole. Merci madame la présidente, monsieur le ministre madame la rapporteure, chers collègues, cet amendement vise à concilier à la fois le sens de l'engagement, mais aussi le respect de la collectivité dans laquelle nous sommes élus, il propose que tout membre du conseil municipal qui sans excuse a manqué 5 séances consécutives cessent d'être membres du conseil municipal, le fait qu'un membre a manqué sans excuses 5 séances consécutives, est constatée par une mention sur le registre destiné à recevoir les procès-verbaux du conseil municipal. En fait, le présent amendement propose d'étendre à l'ensemble du bloc communal commune syndicale Pesci une règle qui existe dans notre République en Alsace et Moselle concernant les démissions en cas d'absentéisme répété d'un conseiller de l'assemblée concernée, article 25 41 9 10 et 11 du CGCT cette disposition serait un moyen de prévenir relativement l'absentéisme répété et non justifiées, d'élus, il est avéré que la pratique des mandats évolue, que l'assiduité a pu diminuer dans le temps, cela a sans doute à voir avec les nouveaux nouvelle forme d'engagement mais aussi à l'évolution des modes de vie, nous connaissons tous des communes dans lesquelles il y a eu un déménagement et Lemaire n'arrive plus à contacter un conseiller municipal, et est ou a nié, ainsi il arrive que des élus quittent leur territoire et ne donne plus signe de vie, empêchant l'arrivée d'un ou compte nouveau conseiller plus motivés, bien sûr, il y a un rapport au civisme dans cette proposition, mais je la présente sous un angle purement technique permettant de fluidifier le fonctionnement dès assemblées locales du bloc communal et je tiens à préciser que je n'ai pas repris une autre disposition du code Alsace qui prévoit de la même manière d'exclure des conseillers municipaux, des conseils municipaux, des conseillers ayant troublé l'ordre qu'ils puissent être exclu pour un temps déterminé ou pour la durée du mandat, je vous remercie.

Le même objet, et même un peu au-delà, parce que pour ma part, je pense également que les procédures d'exclusion, vous savez c'est comme partout. Il y a des règles et quand on enfreint les règles, soit on considère qu'il faut jamais rien dire, soit on prend des décisions, y compris d'exclusion. ça reprend du droit local Alsace Moselle. Il s'avère qu'avant la décentralisation ce ce pouvoir était donc avant les années 80 était dévolu aux préfets, alors on est plus dans la même époque, mais j'ai eu par plusieurs élus des retours et vous aller assez vite comprendre, on peut avoir aujourd'hui des mesures d'obstruction du bon fonctionnement d'une assemblée municipale, dans une commune, quel qu'en soit la taille pour des conflits de personnes pour des majorités, vous pouvez avoir d'un conseiller municipal qui, par exemple, 15 membres, une élection qui se termine à 8 7 et puis une volonté qui peut être durable d'obstruction pour avoir le quorum, premièrement, deuxièmement vous ajoutez dans éventuellement la majorité même si elle fait bloc des modifications liées à des déménagements et vous êtes régulièrement finalement handicapé dans le bon fonctionnement de l'Assemblée, hé bien moi je pense que dans une à un texte de loi sur l'engagement, il faut simplement rappeler que les femmes et les hommes qui s'engage, mais ils font face à leur mandat, faute de quoi ils posent leurs les missions sauf parce que vous avez vu que tout ça est parfaitement organisé et régler en Alsace-Moselle, donc l'idée c'est pas d'être un gendarme, c'est de permettre le bon fonctionnement des assemblées par rapport au fait que, premièrement, les élus sollicitent la confiance de leurs concitoyens, deuxièmement l'obtienne hé ben quand on a la confiance pour 6 ans, on se doit d'être à la hauteur de la confiance que témoigner c'est pas davantage que ça, mais je peux vous dire que dans quelques cas particuliers, ils sont pas très nombreuses, j'ai, j'ai eu le retour mois de d'une des 2 assemblées des maires, on m'a expliqué que finalement il y avait assez peu de recours ou de décisions de ce type, mais ça permet de dénouer assez simplement des solutions de conflit. Merci monsieur Huchon Madame la rapporteure, avis de la commission sur ces amendements. Merci madame la présidente, ces 2 amendements pose une question qui, effectivement, comme l'a dit notre collègue Huchon mais aussi notre collègue Jacques peut créer des situations difficiles, un conseil municipal qui, si je puis dire, brille par son absence, et peut causer un certain nombre de difficultés, donc c'est un vrai sujet en même temps j'attire l'attention sur le fait que les maires ne sont pas toujours avide de constater que, il y a des absences d'un certain nombre de conseillers municipaux qui pourrait conduire, si ce nombre est important à renouveler un conseil municipal, donc c'est un sujet, je répondrai à Monsieur Jacquin que d'une pas il existe déjà des dispositions alors qu'ils sont constatées par le juge administratif, qui peut déclarer un conseiller municipal démissionnaire parce que il est complètement absent en monsieur Huchon, vous faites référence à un droit local qui s'applique en Alsace Moselle qui est antérieur à la constitution et qui effectivement défini des règles définies des règles très précises, vous les avez évoqués, puisque ces dispositions peuvent permettent d'exclure du conseil municipal des conseillers qui ont manqué sans excuse suffisante 3 séances successives ou ayant troublé lors du conseil, il prévoit par ailleurs la cessation des fonctions pour les conseillers ayant manqué 5 séances consécutives, donc je pense que c'est sans doute une vraie question, mais difficile à régler, dont il faut mesurer dont il faut mesurer les les conséquences, sachant qu'on a peut-être eu ce mandat des difficultés particulières, notamment avec l'obligation de constitution de listes à partir de 2000 habitants, les personnes qui s'engager pour Fernand ne mesurait pas forcément l'importance de leur engagement, et on a aussi aujourd'hui des municipaux qui, pour des raisons professionnelles sont amenés à être un peu plus mobile et sont moins disponible, donc la commission a émis un avis défavorable à titre personnel j'émettrai un avis de sagesse parce qu'il y a un vrai débat autour de ça. Monsieur le ministre, vous avez la parole pour la vie du gouvernement. Oui merci madame la présidente, on va reprendre les 2 amendements si vous en êtes d'accord. Dans l'ordre, moi je suis convaincu par l'opportunité du débat que vous portez l'un et l'autre c'est compliqué d'avoir un texte sur l'engagement et au bout d'un moment, de ne pas regarder aussi droit dans les yeux, la situation dans lequel il y a un défaut d'engagement d'ailleurs, à chaque fois dans vos 2 exposés d'émeutes. Qui fait dans vos 2 dispositifs juridiques, vous prévoyez très clairement la situation dans lequel, en plus, les absences sont consécutives et non justifiées. Je sens que ça suscite en tout cas un débat au sein de la commission, en ce moment même. Pardon, monsieur le sénateur. Non, puisque je n'ai pas de débat avec moi-même, au moment où je vous parle en tout cas pas débat suffisamment sonore pour inonder l'ensemble des bancs alentour. Non, de 2 choses l'une, puisque j'étais en train de regarder le dispositif juridique, monsieur le sénateur Husson, il y a juste un mot, enfin il a y a 2 choses dans votre amendement fait droit il y a des absences de 5 séances consécutives, très bien, je pense. Voilà, mais il y a une formule qui pourrait fragiliser peut-être le dispositif vous dites ou conseiller municipal qui sans excuse suffisante, a manqué 3 séances successives du Conseil très bien. L je lis quand même au débat et à l'examen du Sénat et la commission des lois si elle m'écoute ou qui a troublé l'ordre à plusieurs reprises, sans tenir compte des investissements des donc l'un dans un autre registre, on est plus dans le registre de l'absentéisme, mais dans le registre du comportement, au conseil municipal au conseil communautaire format dans une assemblée, je veux juste après peut-être entend le sénateur sont sur le le la. Paternité vous avait la patate et d'amendements sur ce que vous vouliez faire parce que typiquement, là on est de nouveau face à un problème plus démocratique, bien évidemment, y compris d'ailleurs dans cet hémicycle quand quelqu'un proteste énergiquement contre quelque chose, où est la appréciation de la délibération oui la sénatrice Cukierman aurait du souci à se faire bon donc pour toutes ces raisons, je vous propose soit de retirer votre amendement au bénéfice de l'amendement 907 rectifié bis qui pour le coup, lui, est bavard juridiquement parce qu'il prévoit toutes les quatre situations d'appel devant les juridictions administratives, ce qui est à des avantages, donc pourquoi pas, soit de le sous-amender mais ça pour le coup, vous le verrez, monsieur le sénateur sont en enlevant toute cette partie sur le comportement et en ne gardant que l'absentéisme, bon, ça n'a l'air de rien, il est 21 heures 45 et on va introduire en droit, quelque chose qui n'a jamais existé auparavant, qui est de dire que un élu qui s'absente 5 fois consécutives du conseil municipal se verra déchu. De son mandat électif, par décision du maire, votée par le conseil municipal avec potentiellement derrière différents recours c'est pas que neutre, mais une fois de plus, non, mais justement j'en fait exprès, monsieur sénateur pour vous puissiez bien expliqué pour l'ensemble du Sénat au moment où on va voter cette disposition parce que c'est quelque chose de nouveau mot qu'elle le suis favorable puisqu'une fois de plus c'est compliqué d'avoir un test, un texte sur l'engagement sans pour autant à un moment donné, sanctionné, c'est déjà ceux qui occupent des postes et qui ne permettent pas à d'autres suivant de liste, etc, de siéger à leur place, donc c'est un beau débat, je pense qu'il faut la voir donc avis favorable, moyennant le point que je viens d'évoquer. Très bien, merci Monsieur le Ministre, alors. On va peut-être s'occuper d'abord du sort de l'amendement 907 rectifié bis et ensuite on reviendra sur la position de monsieur sont sur son amendement qui fait l'objet d'un avis défavorable de la commission et d'une demande du ministre si à vif avait enfin avis favorable si sous-amendement, mais on le verra dans un second temps, donc on va commencer par le commencement, et je vous propose, s'il n'y a pas de demande d'explication de vote de procéder au vote sur le 9107.

cet amendement ne prévoit pas cette disposition uniquement pour le conseil municipal, il prévoit bien pour l'ensemble des collectivités du bloc communal, ce qui vaudrait dans les communes vaudrait aussi dans les interco ou délaissant dans les syndicats, pas au Sénat, ni au département ni à la région, je tiens à le préciser, madame la rapporteure, vous avez précisé qu'effectivement dans le droit actuel, il faut faire recours au juge administratif, ça prend un certain temps, vous n'êtes pas sans le savoir, moi je pense maintenir cet amendement, il pourrait être approfondie pendant la la navette, c'est effectivement un texte sur l'engagement, j'avais pris soin parce que ça a été travaillé avec mon association des maires de retirer l'aspect trouble à l'ordre qui me semble poser des questions doivent d'opportunités absolument voilà donc je maintiens cet amendement. Alors Monsieur Europe puis après peut-être Madame Gatel répondre à l'ensemble des orateurs. Oui, madame la présidente, tout à fait d'accord sur le fond de ces amendements, moyennant quelques remarques qui ont été faites, notamment sur le trouble à l'ordre public, mais simplement je suis interpellé par la notion d'excuses, c'est à dire où est-ce qu'on défini la notion d'excuses est-ce que c'est dans le règlement intérieur du conseil municipal, est ce que c'est par par une disposition décret parce qu'il a pas mal de jurisprudence sur les excuses qui ont troublé les débats dans un dans dans le tribunal administratif et au Conseil d'État parfois donc je, je pense que la notion d'excuses, nécessite des précisions.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, en qualité de sénateur alsacien je je voterai ces 2 amendements sans faire de détail pour 2 raisons : la première c'est que c'est vraiment tout à fait exceptionnel, mes chers collègues, que quelqu'un ici se puisse se prévaloir du droit local alsacien mosellan pour demander son extension à l'ensemble du territoire national ça mérite d'être marqué d'une Pierre blanche, vous avez compris que je ne veux pas faire la fine bouche et alors la 2ème raison c'est que il est tout aussi rare de voir le Membre du gouvernement, donné un avis favorable, même si ça ne concerne que l'un de ces amendements, donc vraiment merci à mes collègues d'avoir déposé ces amendements et si nous pouvions avoir une belle majorité sur cette extension j'en serai le plus ravie, je souhaiterais d'ailleurs que cela puisse servir à d'autres occasions, puisque mes chers collègues, comme a pu le constater, la commission des lois dans un petit séminaire que monsieur le président de la commission des Lois avait bien voulu organiser et qui avait été particulièrement suivi le droit local alsacien Rouslan a beaucoup d'intérêt, beaucoup d'atouts, quelques inconvénients de temps en temps, mais beaucoup d'atouts, tout particulièrement pour les collectivités locales, mais aussi pour d'autres secteurs qui n'attendent qu'une extension pour effectivement prospéré à l'heure où il faut bien le dire, nous avons une décision du Conseil constitutionnel, qui nous empêche de faire évoluer notre notre droit local autrement que dans un sens du rapprochement avec le droit général, là pour le coup, c'est juste l'inverse qui est en train de se passer et je suis ravi.

qui introduit la possibilité pour l'assemblée d'apprécier et moi ce qui me gêne dans l'amendement de monsieur Jack hein c'est que on, on s'en remet au tribunal administratif, je croyais que nous étions dans une logique d'engagement, de proximité et de simplification, je trouve que telle qu'il est rédigé Monsieur Jacquin, je dis pas que c'est votre intention, mais ça m'inquiète un peu, de se dire que le conflit ou les difficultés entre des collègues élus va se régler devant le tribunal administratif, moi je trouve que l'amendement de monsieur Huchon est beaucoup plus intéressant parce qu'il renvoie la responsabilité des collectivités territoriales et donc je ne voterai sûrement pas l'amendement de monsieur Jacquin et je me propose de voter l'amendement de monsieur sont parce que c'est un amendement de liberté de responsabilité. Merci monsieur Delage Madame la rapporteure, vous avez la parole. Merci madame la présidente, donc on voit bien que ce débat, ce débat et nourri les sans doute justifié, moi j'ai dit à titre personnel, sagesse, avec les réserves que j'ai mis dire hein, s'il y a un caractère automatique, il faut veiller à ne pas mettre en difficulté des municipalités qui verraient leur nombre obligatoire de conseillers municipaux disparaître et qui contraindrait ces municipalités à refaire des élections générales, deuxièmement, je suis assez sensible à l'argument qui a été évoqué sur la nature des absences qui pourraient être prises en considération, on imagine un congé maternité, un accident de voiture ou que sais-je, ou une contrainte professionnelle qui fait que le conseiller municipal est empêché, donc le débat, il a raison d'être maintenant moi j'attire l'attention sur les effets collatéraux qui peuvent se produire, y compris le plus redoutable d'entre eux qui est celui d'une obligation de renouvellement du conseil municipal. Merci madame la rapporteure monsieur mise, on a demandé la parole pour explication de vote. Merci madame la présidente, 8 je voudrais rassurer ceux de mes collègues qui ne le seraient pas avec cet amendement, que ce soit celui de monsieur Hue 100 ou même celui de Monsieur Jacquat, nous n'allons pas à l'aventure, c'est un dispositif qui existe, qui a fait ses preuves et qui est efficace, je l'ai moi-même expérimenté, mais je peux vous dire que ça exprime auprès des autres conseillers municipaux une une une un rappel au règlement, quand on s'engage quand on a l'honneur d'être élu par sa commune sa ville, hé bien on a des engagements, et c'est une bonne manière de le rappeler, je rappelle que 5 absences consécutives sans excuse aucune ça justifie qu'on réagisse. transposons cette règle à une assemblée parlementaire, ne prenons pas le Sénat, bien sûr, mais par exemple, l'Assemblée nationale, vous jugeriez légitime que la première sanction à laquelle on pense soit l'exclusion définitive, je trouve que c'est un peu raide, je pense qu'il faudrait concevoir les choses avec davantage de gradation que la piste qui est assez ouverte, c'est une piste qui mérite d'être explorée mais en ce qui me concerne, après l'avis de sagesse qui a été émis, je dois vous dire que je trouve que ça va un peu vite et que ça peut ensuite être recyclés dans des conflits politiques locaux ou on discutera des excuses avancées par quelqu'un qui aurait eu un accident de voiture, une maternité qui aurait manqué 5 conseils municipaux ou un déplacement professionnel de longue durée à l'étranger et on dira bonne ton excuse n'est pas légitime, tu es viré, dans certains cas au fond appliqué de bonne foi, cette règle pourrait être justifié mais j'aimerais mieux qu'on puisse avoir une modulation des sanctions, une hiérarchie de sanction et qu'on n'aille pas directement aux extrêmes, alors que c'est quand même des élus du suffrage universel et que, quelle que soit la taille de la collectivité dans laquelle on est élu, hé bien le lien entre le citoyen et son représentant est le même, on a été envoyé dans une assemblée, par la volonté du suffrage universel, on doit pas pouvoir en être exclu par une délibération de son assemblée, voilà la raison pour laquelle moi je voterai contre. Merci monsieur le président, j'ai encore 2 demandes d'explications de vote Monsieur Bigot, vous avez la parole. Et de tout sont

alsacien mosellan et président de la commission droits de devoir local a actuellement après lui de de cette aspiration alsacienne, ceci étant, le texte très peu utilisé en Alsace et effectivement, c'est le conseil municipal qui décide si la personne cesse ses fonctions il y a pas d'automaticité, ce qui paraît sage et c'est la raison pour laquelle ce texte n'est pas souvent appliquée mais il est, il y a d'ailleurs une décision récente du une grande ministre sera-t-il de Strasbourg qui a confirmé la décision d'un conseil municipal et je dois dire que dans la situation actuelle où on constate de plus en plus d'absence, moi j'ai été maire pendant 20 ans dans le 1er mandat, je n'avais jamais d'absence dans le second mandat, je n'avais jamais d'absence dans le 3ème, j'ai commencé à noter et on en a de plus en plus et donc je pense que rappeler, comme l'a dit notre collègue les collègues vont devoir dire c'est pas automatique et puis à la d'autres sur la liste qui peuvent venir être élu, ça paraît bon, mais il faut que faut peut-être amendé le texte en précisant que c'est sur délibération du conseil municipal, c'est-à-dire qu'il y a pas d'automaticité, parce que les circonstances peuvent faire culte.

je pense en effet qu'il y a un vrai, un vrai problème parce que quand on est conseiller municipal, on est censé avoir un engagement dans le dans le temps. ça pose un bon problème vous savez que la question de l'absentéisme et dans dans beaucoup d'instances des collectivités locales, c'est vrai dans le département, c'est vrai dans les régions, certaines régions ont mis des règlements en place à dessein, ce qui me gêne, ici, c'est un peu l'automaticité après 5 absence c'est vrai que c'est un engagement mais l'automaticité peut faire en sorte que à priori, ça peut poser des difficultés et ça peut donner lieu aussi à des règlements de comptes politiques éventuellement une modulation me semblerait de de bon aloi, sachant que, pour reprendre l'image de Monsieur, le président de la commission des lois, il est évident que c'est difficile d'imposer à d'autres, c'est-à-dire aux conseillers municipaux, des règles plus strictes que celles qui s'appliquent aux arènes parlementaire et je pense pas qu'il faille faire 2 poids 2 mesures, on peut faire des modulations, on peut faire des règlements, mais il me semble que l'automaticité en l'espèce, me pose problème. alors. D'abord, monsieur le ministre a demandé la part. Les explications oui, madame la présidente, je me remettrai à la à la sagesse du Sénat juste pour peut-être lever une inquiétude, telle qu'elle a été évoquée : le caractère de la justification, ce qui permettra de se justifier et bien évidemment, je ne sais pas comment le sénateur Husson compte sous-amender son amendement s'il compte le sous-amender le maintenir mais peut renvoyer à un décret, voire même un décret en Conseil d'État si vous pensez qu'il faut y consacrer la force qu'il va bien, dans lequel endroit nous ne manquons pas de référence dans le droit du travail et autres, dans lequel on peut lister ce qui fait l'objet pour répondre aux sénateurs Rapin et à sa juste remarque lister les choses un certificat médical, que sais-je, enfin voilà, donc il faut bien cumuler les choses dans l'esprit du sénateur Husson c'est faux, que ce soit consécutifs, il faut que ça soit du justifier un renvoi un décret peut le faire faut enlever bien évidemment la question des troubles après se posera la question entre nous sur ce dispositif. Du caractère constitutionnel ou pas de cela, puisque ce qui a été confiée par le suffrage universel est toujours délicat à retirer, c'est aussi pour ça que l'inspiration du droit alsacien, monsieur le sénateur est moins évident mais, comme le président bat depuis la semaine dernière m'invite à être aventurier sur le terrain de la Constitution, puisque le sénateur président ministre bah m'invite à faire preuve d'audace sur le terrain du droit et savoir entendre qu'il faut une volonté politique pour parfois pousser un peu les limites du droit, moi, je m'incline devant la sagesse du président bah, et donc si vous pensez qu'on peut tenter cette aventure, on peut la regarder, on peut essayer de la de la peut-être de la parfaire un tout petit peu, dans le cas de la navette est allé parce qu'on est pas prêt afin d'importe quoi parce que c'est quelque chose de grave si on sent d'ici là, la parce que, blague à part, je suis assez d'accord avec ce président de la commission des lois a indiqué si d'ici à la fin de du débat parlementaire, on voit qu'on n'arrive pas à accoucher d'un dispositif complètement stabilisée sur le terrain juridique propre qui évite toute forme de récupération politique politicienne dans des cas qui nous ferait pas plaisir, hé ben on le retirera du texte d'un commun accord, tous ensemble, en tout cas je comprends que vous ayez envie d'interroger la notion de responsabilité parce que ce n'est pas démagogique poser cette question et c'est assez noble, parce qu'une fois de plus, on parle de crise de l'engagement de celles et ceux qu'on a du mal à trouver pour occuper des postes mais aussi celles et ceux qui auraient bien aimé les occuper et avec certains qui ne siègent pas, qui par définition empêchent d'autres de s'engager à leur place, et donc c'est aussi une manière de répondre à la crise de l'engagement, donc je vous propose cette voie de sagesse. C'est chez ces. Merci monsieur le ministre, madame, merci, vous avez la parole. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je voudrais soumettre à votre réflexion, un cas pratique que j'ai eu dans ma commune, d'une confirme municipal qui a développé un cancer du sein et qui n'a jamais voulu que ce soit connu, moi seul à l'époque j'étais maire savait pourquoi elle ne pouvaient assister aux séances du conseil municipal, c'était un lien de confiance qu'il y avait entre nous et j'ai expliqué aux conseillers municipaux, elle ne sera pas là point donc je crois que cette notion d'automaticité ne doit pas s'appliquer, mais qu'il y a une notion de confiance et elle ne voulait pas qu'on sache qu'elle était malade, ce n'était pas public, c'était un secret entre elle Merci, cher collègue, alors je vous propose maintenant que nous procédions au vote sur ce premier amendement alors. Qui est pour. Normalement, si je respecte le règlement à partir du moment où les explications ont eu lieu sur un amendement et sur cet amendement, les explications de vote ont eu lieu normalement, on peut plus sous-amendé, c'est que le sous-amendement Servent les explications de vote. le règlement c'est ça. On applique le règlement on l'applique pas. Donc on va procéder au vote. Donc, je vous propose de procéder revote qui est pour. L'amendement le premier amendement, c'est-à-dire le 907 rectifié bis. Qui est contres. Qui s'abstient. L'amendement n'est pas adopté. Alors maintenant, nous allons commencer par Monsieur, qui va prendre la parole. Suite à la question qui lui a été posée par monsieur le ministre, sur. Les et les modifications potentielles de de son amendement. Voilà, merci, merci à la présidente, moi je propose effectivement de rentrer dans le sous-amendement, je vais le proposer et de faire prospérer le travail parlementaire, la navette et je souscris, monsieur le ministre, à tout ce que vous avez dit, y compris ici pour des raisons je dirais juridiques, enfin etc, il faut pouvoir atterrir je dirais tranquillement et intelligemment parce que je veux, je veux dire quand même rappeler 2 ou 3 éléments : premièrement, c'est des sujets qui m'ont été qui ont été soulevées lors de rencontre que j'ai eue avec plusieurs maires de mon département, donc je vais pas raconter l'histoire, mais c'est quand même la première chose la 2ème moi j'entends, je vous remercie les, les, les, les élus d'Alsace Moselle vous dites c'est bien tout ce qu'ils peuvent faire prospérer le droit local ou s'en inspirer, je vous invite aussi dans ce cas-là, ne l'oubliez pas honte le à la réciprocité, ce qui est vrai dans un sens, c'est aussi vrai dans l'autre, quand il y a des bonnes solutions, troisièmement, que je sache, et ça a bien été rappelé par notre collègue en Alsace Moselle, ça arrive rarement. Les élus ne sont pas plus hors-loi. C'est des dispositions législatives, donc je je propose maintenant de sous-amendé dans le deuxièmement donc en supprimant effectivement tout ce qui touche à ordre public puisque c'est moi factuel, il y a une appréciation, on peut même supprimé sans excuse. Enlevez le suffisante parce que comme ça, y a pas d'appréciation, on est dans le parallélisme des formes, on dit bien sans excuse et donc pour ma collègue Madame Mercier compte il y a simplement une information qui est donnée par une élue et porté par un homme, le maire, enfin pour moi, la personne est excusé, on lui demande pas de justifier de dire bon, et puis comme l'a dit le ministre, on verra le décret etc c'est juste d'apporter du bon sens du respect de l'engagement, etc, et je rappelle enfin que, pour l'exclusion il faut aucune excuse pendant 5 séances consécutives, ce qui veut dire que, parfois, c'est plus d'une année. Dans certaines communes, voilà donc il y a pas de chasse aux sorcières, il y a simplement, je crois que ça a été dit, le respect des engagements qui sont pris, y compris devant le suffrage universel. Huchon donc avant d'ouvrir les explications de vote, je veux bien être certaine d'avoir bien qu'on. Oui, l'amendement rectifié je vais relire en tout cas la partie qui est réécrite, qui est donc se sont ajoutés 2 articles ainsi rédigés article, elle vend 200 212 1 tout conseiller municipal qui. Sans excuses a manqué 3 séances successives du Conseil.

peut, par décision de l'Assemblée, être exclus du conseil municipal pour un temps déterminé ou pour toute la durée de son mandat, quant à l'article suivant le le par grâce suivant, on n'y touche pas, on est bien d'accord.

c'est donc sur cet amendement rectifié, que nous allons écouter les explications de vote et s'il n'y a pas d'explication de vote on procède. Au vote le prix. Monsieur le président, ben, vous avez la parole. Oui je je salue les corps de notre collègue Jean-François Husson, mais j'ai besoin de comprendre qu'est ce que c'est qu'une excuse.

Il n'a pas la parole, le sens de ma question, c'est de dire que cette disposition ne peut avoir aucun effet pratique parce que le conseiller municipal absent, il lui suffira de dire je ne, je ne suis pas là vendredi prochain, c'est une excuse, oui, mais alors à ce moment-là, pourquoi légiférer parce que le la disposition qui permettrait d'exclure un conseiller municipal qui est régulièrement absents serait immédiatement privé de tout effet parce qu'il aurait présenté une excuse, c'est-à-dire je ne peux pas être là vendredi prochain. Président Monsieur Jacquin, vous avez la parole. je respecte pleinement vos décisions, j'ai pas trop compris comment vous avez animé la séance pour faire en sorte que je m'exprime avant Monsieur Husson, alors que c'était les 2 mais c'est pas grave, je vais être constructif madame mon amendement n'est plus, et je vous rapporter dès des précisions sur celui-ci, je proposerai que le sous-amendement soit complété au bloc communal et pas uniquement au conseil municipal, c'était une différence importante entre nos 2 amendements et ensuite, je pense, c'est important de voter cet amendement pour qu'effectivement dans la navette qui puisse être éventuellement améliorer et corriger ça me semble être une disposition constructives sur un texte qui porte sur l'engagement et quand on parle de 5 absences injustifiées, c'est des cas rares et prolongé, ce ne sont pas des chasses aux sorcières donc quelqu'un qui viendrait à ne pas dire je ne suis pas là parce que j'ai piscine, hé bien ils seraient concernés, ça arrive maintenant, des gens qui perdent leur attache locale ne donne plus aucun signe de vie, ces, ces gens-là que nous visons dans cet amendement. Monsieur Jacquin. Pour vous redire quelle est la règle Monsieur Jacquin, quand nous avons des amendements en discussion commune, on est, on les présente successivement, on a un avis de de la rapport. Sur un avis du ministre sur chacun mais ensuite on procède au vote un par un et donc les explications de vote, on commence par le premier amendement et ensuite on passe aux explications de vote sur le second amendement et donc on le fait en 2 temps et c'est pour cela qu'effectivement Monsieur Husson a répondu dans un second temps, à la proposition du ministre, voilà ce qui a valu, effectivement, cette organisation alors je cède maintenant la parole à monsieur Madame la présidente, monsieur le Ministre, chers collègues, je suis bourguignon et fils de Laurent, né à Forbach et je pense qu'il y a pas d'excuses s'excuser, a proposé tels amendements que j'ai cosigné en 4ème position parce que notre collègue Husson a parlé du mot respect. Et l'Alsace et la Lorraine, c'est un territoire de respect en général peu de gens ont besoin de s'excuser parce qu'il ne manquent pas, mais j'aimerais que cet avènement qui soit accepté ou pas, je voterai pour cet amendement qu'il fasse, qu'il agisse par capillarité ou par porosité pour que le respect règne sur tout le pays, merci. La parole est à Monsieur Detraigne. Merci madame la présidente, si je comprends bien, nous gardons l'article L de 21 21 tout conseiller municipal qui sans excuse suffisante, a manqué 300 successives du Conseil n'en peut, par décision. Bon ok, peut, par décision de l'Assemblée, être exclus du conseil municipal pour un temps déterminé ou pour toute la durée du mandat en fait le peut me gêne parce que ça veut dire que c'est la tête du client.

Monsieur le Ministre, mes chers collègues, il me semble que la moindre des choses, dans nos conseils municipaux, c'est le respect et c'est le respect également des présence l'assiduité quand même un petit peu et je pense que la moindre des choses quand on est absent, c'est de dire de d'envoyer un petit mot ou d'appeler le maire ou un conseiller municipal ou un adjoint en disant voilà, je ne serais pas là, c'est ça une excuse, on demande pas de savoir si la personne à Tahiti ou si elle a un vrai problème de fond, il me semble que la moindre des choses, c'est quand même de s'excuser et souvent dans nos conseils municipaux, on a des gens qui s'inscrivent qui se font élire et qu'on ne voit pratiquement plus et ces gens-là, il faut qu'il comprenne en amont que maintenant, ce ne sera plus possible, et il me semble que cet amendement va dans le bon sens, et personnellement je le voterai. Merci, la parole est à monsieur Bockel. J'interviens un peu dans le sens de de Alain Houpert en en soutien de l'amendement je pense je pense intelligemment, sous-amendé de de Monsieur Husson, parce que bien sûr, je comprends ce que dit monsieur sur la notion d'excuses et il a raison, mais le simple fait que cette règle existe si peu contraignante soit-elle, avec tous les éléments de respect qui ont été rappelés par d'aucuns, c'est un élément soit qui est connu, qui peut être d'ailleurs dans certains cas, repris quand il y en a un dans le règlement intérieur et, à partir du moment où une règle est connue, ne pas l'appliquer. C'est déjà en soi dans le collectif du Conseil une difficulté un problème ça amène à échanger et à dialoguer et quelqu'un qui serait ou qui auraient le sentiment, comme vient de le dire Monsieur de traîner un moment donné, d'être peut-être victime de ne pas plaire etc, hé ben, il suffit de venir ou alors de préciser les choses aurais je peux vraiment pas venir et l'excuse peut être précisée, le cas échéant, mais on en aucun cas on est soumis au vote du conseil en vue d'une sanction éventuelle de manière subreptice, donc je pense que la perfection n'est pas de ce monde et et vouloir avoir une notion d'excuses qui nous sécurise absolument pense que au fond ça ne va pas un très grand intérêt, je pense que voter cet amendement ainsi sous-amendé, avec les navettes et tout ce qu'a dit le ministe tout à l'heure sur des éventuels sécurisation réglementaire, je pense que c'est un progrès et c'est un message qu'on fait passer et c'est pas si mal.

les Alsaciens Mosellans ne sont pas non plus parfait, il faut être très clair les poudres, décision que nous avons la dernière en date, abstraction de Strasbourg méritent d'être examinés, parce qu'effectivement, elle témoigne pour répondre à Monsieur Detraigne que il y a d'abord une motivation de la délibération du conseil et que cette motivation, fait l'objet d'un contrôle du du juge administratif, qui ne peut pas y avoir d'excès de pouvoir à l'égard de la décision de l'un des membres et sur la nation d'excuse suffisante mais bien évidemment il appartiendra juridiction de vérifier c'est bien motivé, donc je crois qu'il y a quand même un entourage et qui peut être encore affiner, comme l'a dit Monsieur le Ministre, je pense que ça mérite que on ne vote cet amendement. si on rentre dans des procédures d'hyper jeudi dit il arrive à Sion pour, à l'issue, savoir si finalement au départ, le conseil municipal avait tort, avait raison de suspendre et pendant ce temps-là, qu'est ce qui se passe quant au remplaçant ou pas, je pense que c'est vite ingérable très précisément ce qui est écrit, puisque cet amendement et donc cet article, s'il était ainsi voter s'appliquera bien évidemment à toutes les tailles de communes, moi je crois que ça peut-être faire sourire ou choqués, quoique notre collègue Détraigne dit que c'est à la tête du client, mais inévitablement le fait majoritaire existant quand même dans les communes à scrutin liste au-delà de 1000 dès lors qu'on fait voter par le conseil municipal, on peut envisager parce que je veux bien qu'on soit dans un monde des bisounours sous la grande famille des élus locaux, tout se passe très bien et qui aurait jamais de soucis nulle part, mais parfois c'est dans les repas de famille que les discussions sont les plus violentes et que donc je crois que, qui va de retenir. Le la notion d'excuses qui va présenter l'acceptation de l'excuse et quel va être le vote. Kim, à un moment donné, sera celui d'un fait majoritaire dans un cas comme dans l'autre, quelle que soit finalement celui qui est maire de de la commune concernée et donc autant j'entends le le souci qui est de donner de l'exemplarité mais vous savez, quand on a commencé à mettre le doigt sur les questions de transparence, on peut toujours laver plus blanc que blanc, ça ne suffit pas, donc je crois qu'est ce qu'on est sur un vrai texte qui veut redonner l'engagement, la proximité et la responsabilité des élus ou faire sous-entendre finalement ici que on a parlé pendant plus d'une heure de comment est-ce que l'on sanctionnerait effectivement quelques brebis galeuses qui existent et qui ne participe pas aux travaux municipaux dans la commune dans laquelle ils ont été élus, je crois qu'il faut aussi faire attention à cela et nous ne voterons pas cet amendement même sous-amendé. Merci Madame Tucker même nous avons encore six demande de prise de parole, donc nous commençons par monsieur Lafont. Madame la présidente, sous cette appellation, je serai donc bref pour pour souligner que d'abord ce cet amendement manifestement France fait débat, moi ce qui me pose problème, c'est une forme de rigidité dans la rédaction de l'amendement qui laisse à penser d'abord qu'il y a un problème massif de de d'absentéisme dans les conseils municipaux, alors que généralement c'est quelque chose qui est assez marginal et qui, et qui résulte de quelques cas très particulier qu'il vaut mieux traiter de façon proportionnée et adaptée, plutôt que d'en faire une règle générale c'est possible dans le règlement intérieur de prévoir un certain nombre de de dispositions et de le faire de manière souple et intelligente, à mon avis peut être fait sans qu'on ait besoin de légiférer là-dessus. Si Monsieur Lafond la parole est à monsieur Alizart. Oui, madame le président, monsieur le Ministre, moi je ne vous cache pas que cet amendement me dérange un petit peu dans sa conception, tout simplement parce que j'avais cru comprendre, nous étions sur un texte à la base d'origine sénatoriale, repris par le gouvernement, et c'est un texte qui, finalement, veut donner de la souplesse de la liberté et on réglementé on réglemente je été maire pendant 22 ans mais comme plein de gens ici dans cet hémicycle, j'ai eu effectivement à subir de l'absentéisme dans mon conseil municipal des gens de la majorité des gens de l'opposition, j'aurais tendance à vous dire que si sanction il doit y avoir, elle doit venir des électeurs lors de l'élection suivante, donc je suis pas particulièrement favorable à cet amendement, y compris sous-amendé qui risque d'ailleurs de générer des règlements de compte dont on n'a pas forcément besoin, dans nos conseils municipaux. Madame la. Présidente, monsieur le ministre, je voudrais tout d'abord à rappeler que il n'y a aucun caractère d'automaticité dans ces exclusions aucun caractère d'automaticité, j'insiste là-dessus, il faut tout d'abord que la proposition d'exclusion faite par le maire soit bel et bien inscrit à l'ordre du jour du conseil municipal et par conséquent, figurait sur la convocation s'occupe, je parle là ce qui se passe en droit local puisque j'ai l'occasion de pratiquer cette exclusion, donc l'intéressé a tout à fait la possibilité de venir s'expliquer ensuite, s'agissant d'une délibération du conseil municipal, elle peut bien entendu être déféré au tribunal administratif. Aussi bien par le préfet que par l'intéressé, s'il n'est pas satisfaite de son exclusion. Donc des droits de la défense ne paraissent tout à fait garanti, ensuite je voudrais préciser que j'étais président des maires du Haut-Rhin pendant 22 ans, et j'ai eu l'occasion de constater que ces dispositions d'exclusion ont effectivement était très peu utilisé et pourquoi elles sont très peu utilisés ben tout simplement parce qu'elles ont un pouvoir dissuasif tout simplement et ça pouvoir dissuasif vont donc aussi bien pour les abstentions au conseil municipal, que ce qui se cache derrière, ça veut dire l'abstention aux réunions des commissions et des groupes de travail parce qu'en général, ceux qui s'abstiennent absolument tout. Alors en ce qui concerne l'atteinte à la liberté de l'élit municipal argument que maintenant arrivé de lire et d'entendre la liberté du conseiller de participer en au travail du conseil municipal, je rappelle que l'élu a toujours la possibilité de démissionner et de céder la place au suivant de la liste, puisque maintenant à des listes à partir de 1000 habitants ce qui clarifie la situation, il ne semble il n'est pas raisonnable de permettre à certains d'être absent à leur guise selon leur envie mais de réapparaître, et comme par enchantement dans les mois qui précèdent les élections municipales à venir et de se mettre à critiquer sévèrement le travail des colistiers qui eux ont sacrifié une partie de leur vie familiale, voire professionnelle pour le bien commun, c'est pourquoi je voterai cet amendement. Oui, madame la présidente, messieurs les rapporteurs et présidents, monsieur le ministre, comme ça a été rappelé, comme beaucoup d'entre vous, j'ai été maire. au cours de mandat, il y a un élu du conseil municipal, que je n'ai pas revu de jusqu'à la fin du mandat, ça a duré de 3 ans. Mais, de par les textes, même s'ils ne venaient jamais, j'ai été contraint de le convoquer à chaque réunion du conseil municipal et s'il était exclu, ça m'aurait évité au moins d'avoir le convoquer sur toutes les instances, ce dont il était membre, ça a le mérite d'être clair, c'est pour ça que je voterai cet amendement. Merci messieurs Lluch la parole est à Madame Tetuanui. Oui. Oui merci madame la présidente. J'ai écouté mes collègues aurait beaucoup d'argent sur depuis quelques jours

quand nous sommes élus dans les conseils municipaux et c'est le peuple quand même car décidé de nous envoyer et et prendre des mandats, il y a des dispositions actuelles non mais monter ça

ou bien comment vous voulez aller faire appliquer ça on Polynésie Polynésie-Française enfin, pour ceux qui connaissent un peu.

pour les élus de l'autre commune pour venir au conseil municipal, partant de mer calme, bon ce car le mal de mes chers collègues n'y allait pas, c'est pas la paix.

L'Alsace revient. Oui, même à la présidente, monsieur le mise, mes chers collègues, je ne connais naturellement pas la situation de la Polynésie et je ne prétends pas répondre à notre collègue, mais vu la tournure de de ce débat, permettez-moi juste de faire une rapide mise au point, j'entends naturellement et les critiques qui ont été formulées sur la rigidité du système sur peut-être une certaine atteinte aux libertés des uns et des autres, la difficulté de mise en oeuvre, mais permettez-moi juste de vous rappeler que ce texte est appliquée et applicable en Alsace depuis des décennies, et il n'a jamais posé le moindre problème, comme l'on dit tous mes collègues alsaciens, il n'en pose pas parce qu'effectivement il est appliqué avec souplesse et naturellement, comme ça a été dit tout à l'heure, fort justement, toute décision du conseil municipal à l'égard d'un conseiller municipal et soumise, le cas échéant au contrôle du juge administratif. C'est juste un rappel, l'Alsace et pour autant que je sache même intégré au Grand-Est une région française, j'ose dire, une région française, il y a pas de raison que ce qui fonctionne chez nous, ne puisse pas fonctionné ailleurs. Merci, Monsieur Richard, la parole est à monsieur Grand. mais mes chers collègues, moi je suis un peu étonné par cet amendement parce que si vous avez un maire avec qui vous êtes opposé il mettra les conseils municipaux, les mardis et les mercredis, et donc naturellement au choisirez au être ici est comptabilisée par les services, être au Conseil de métro pour à la commune, moi je vois à Montpellier, mais dans les conseils de métropole, c'est toujours le mardi, bon, donc je demande l'indulgence de la présidence pour mes absences éventuellement à venir le mardi, merci. monsieur grand c'est bien noté, alors je crois que nous en avons fini avec les explications de vote, si vous le voulez bien nous allons maintenant passer au vote sur l'amendement 721 rectif. Equateur présenté par Monsieur Husson qui de ce fait, reçoit un avis favorable de la part du ministre et de la part de la Commission, un avis défavorable je mets aux voix l'amendement qui est pour. Qui est contres. Qui s'abstient l'amendement n'est pas adopté. nous passons maintenant, après l'article 11 inquiet-ce un amendement 274 rectifié bis, il est présenté par Monsieur Prince. Merci madame la présidente, j'espère qu'on va aller un peu plus vite dans l'esprit de la loi notre la fusion de syndicats devait permettre d'optimiser le service public, sur l'ensemble des territoires, toutefois, il convient de préciser que cette volonté d'optimisation génère parfois des complications importantes dans sa mise en oeuvre, notamment en raison du mécanisme de représentation substitution en effet tout en incitant à mieux gérer les territoires en regroupant 2 syndicats à compétences identiques, la législation conserve dans le même temps, des mécanismes qui mènent au maintien de la situation antérieure avec des transferts de compétences en cascade, par ailleurs, cette situation n'est pas sans conséquences sur le plan financier ainsi cet amendement, qui se concentre sur les conséquences des fusions de syndicats mixtes propose d'attitude et d'instituer une faculté de retrait du syndicat mixte en question avec l'accord de son organe délibérant. C'est bien, Monsieur le Ministre, même avis madame la présidente, hé bien je vais mettre aux voix cet amendement 274 rectifié bis qui est pour. Qui est contre. S'abstient, il est adopté, après l'article 11 qu'inquiet ce 2 amendements identiques faisant l'objet d'une discussion commune le 340 80 de rectifier, terre, il est présenté par Madame Moret riche. Merci madame la présidente, monsieur le Ministre, mes chers collègues, l'attribution des sièges de conseillers communautaires dans les instances intercommunales est basée sur la population municipale il ne prend pas en compte la population touristique, les communes touristiques ne sont alors que faiblement représentée à l'échelle intercommunale malgré leur abondement financier parfois largement majoritaire, leurs élus perdent alors la maîtrise de projet et politiques impactant directement le développement économique de leur commune, et de ce fait, sa capacité à générer des retombées pour l'ensemble du territoire de l'intercommunalité, afin que les enjeux touristiques ce mieux intégrés dans l'ensemble des décisions prises à l'échelle intercommunale, il pourrait être pertinent de prendre en compte la population DGF au lieu de la population municipale pour leur porte-partition déchets dans l'objectif de disposer d'une évaluation de la situation actuelle et de définir des mesures d'amélioration, il est donc proposé que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur la représentation des communes touristiques dans les instances de décision des intercommunalités. Merci, cher collègue, la parole est maintenant à Madame Bert et pour présenter l'amendement 500 537 rectifié bis. Oui, je vous remercie, madame la présidente, donc mon amendement est défendu, c'est le même j'aimerais toutefois insisté sur l'importance pour les stations particulièrement les stations de ski d'avoir une meilleure représentativité au sein des intercommunalités puisque elle pèse très fortement sur le plan économique dans l'intercommunalité et sont très très peu représentées au regard de leur population résiduelle donc a minima à prendre en compte la population DGF serait très bien, je prends l'exemple par exemple de la communauté de communes de Haute Tarentaise avec des stations de ski que peuvent être Tignes ou Val-d'Isère que sont ces ces grosses stations qui pèse très très peu dans l'intercommunalité et qui n'ont que 2 représentants donc une nécessité de se pencher sur cette question, je vous remercie. aujourd'hui, c'est bien la population municipale qui est prise en compte et pas la population touristique, on a longuement parlé de de de ce critère, un peu bloquant moi j'entends votre préoccupation, vous proposez qu'il soit fait un rapport sur ce sujet, vous connaissez l'appétence du Sénat pour Les les rapports sur un sujet un peu difficile à traiter d'une manière au niveau national, donc c'est une demande de retrait ou à défaut un avis défavorable. Merci, Monsieur le Ministre. D'ailleurs, je note à chaque fois que des différents sénateur montagnard ne sont pas en reste, en amendements et d'ailleurs, le gouvernement et le Parlement accompagne cela avec bienveillance à chaque fois a commencé à faire rentrer la question de la population touristique pour calculer le nombre de sièges de représentation au conseil communautaire c'était en encore pas prendre la population réelle mais prendre la population DGF et à mon avis à faire et à générer des exceptions qui sont absolument redoutable. Deuxièmement, il y aura une difficulté, c'est-à-dire que le touriste seraient comptés 2 fois, une fois dans son lieu de résidence principale, on le contraire dans la représentation démographique dans son ensemble, commune de l'intercommunale de là où il habite et puis on le contrer une 2ème fois, là où a sa résidence secondaire, je le vois comme un amendement d'appel a toujours. Prendre en considération en compte les questions liées aux communes touristiques, néanmoins, une fois de plus dans la représentation politique dans les intercommunalités, ça me paraît très compliqué que de que de rentrer dans cette discussion-là donc : demande de retrait pour les 2 amants. Merci monsieur le ministre, monsieur Loïc Hervé demande la parole pour explication de vote. Merci madame président monsieur Miss, mes chers collègues, sans méconnaître les difficultés que ça pose en termes d'égalité devant le scrutin je voterai cet amendement parce que je constate dans nos territoires de montagne, mais ce pourrait être valable d'ailleurs sur le littoral français, la part de ces communes dans le budget de l'intercommunalité telle que la différence qui existe entre leur puissance économique et leur très faible représentation au sein du conseil communautaire mais je ne parle pas seulement de sous-provenance viendrait, je veux parler autant terme mais qui sont équipés comme telle et ça crée des frustrations légitimes pour les élus de ces collectivités là donc la demande de retrait où l'avis défavorable n'apporte pas une réponse suffisante pour pour que nous puissions renoue retourner vers les élus qui nous pose cette question là qui est une question difficile, nous sommes à 6 mois des élections municipales et nous avons un mal fou à répondent à trouver des correctifs parce que dans la gouvernance de l'intercommunalité,

assez peut-être trop fait, mais au prorata Numéris et là on est dans un cas de figure tout à fait particulier ou ces communes ont un poids économique un poids d'équipements, un poids qui existe dans le territoire qui n'est, qui est sans commune mesure avec leur représentation au sein du conseil communautaire qui est très largement sous-représentées, donc je suis vautré par solidarité avec les collègues qui ont défendu ses qui ont déposé ça amendements et qu'ils ont bien défendu et je le dis, ça concerne les territoires touristiques au sens large du terrain, n'ayez pas en tête que les stations de sports d'hiver parce que je sais tous les fantasmes qui existe autour de ces stations qui sont forcément des paradis sur terre, alors que les mais les élus qui les qui en ont la charge, ont des responsabilités considérables et des moyens souvent beaucoup plus faible qu'on ne l'imagine, mais ça concerne aussi des territoires littoraux ou des territoires touristiques pas dans d'autres Syntec Tour de France, qui est, mes chers collègues dans sans doute qui existe dans votre département. Merci monsieur Hervé, monsieur le ministre, vous avez la parole. Oui, madame la présidente j'entends ce que vous dites, je dis juste que, comme ici, on crée le droit, il faut faire attention à tout ce que l'on peut ouvrir aussi comme brèche puisqu'à ce moment-là, vous êtes maire d'une ville dans lequel vous avez un grand quartier politique de la ville, les politiques urbaines de logement ou de politique de la ville sont au niveau intercommunal et donc les communes parfois plus petites ou rurales ou qui n'ont pas QPV comprennent moins bien également où il y a moins de représentation politique donc pas ce que c'est qu'parce que la politique de la ville est une compétence intercommunale, il faudrait qu'une commune qui a un QPV et une sur-représentation en élus communautaires, les questions de représentation, elles sont, elles, sont éminemment démocratique, elles se sont éminemment égalitaire, c'est pas un hasard si la Constit. Si on dit des choses sur le sujet, et une fois plus, j'entends le besoin d'différenciation pour redire le mot clé du moment, sur lequel on doit tous travailler avancer, mais je doute que ce soit d'ailleurs, un rapport du gouvernement remis au Parlement qui changera beaucoup la donne sur le sujet, la vraie question, c'est comment on arrive à avancer sur la différenciation et je pense, monsieur le sénateur Hervé en tout cas je forme le voeu que ce que nous avons adoptée collectivement sur le pacte de gouvernance au début de la discussion la semaine dernière, permettent d'adapter aussi de bonnes pratiques pour faire en sorte qu'une commune qui a un niveau d'activité ou une nature d'activités spécifiques puissent être intéressé à la gouvernance de manière différente, en tout cas c'est pas par le fait de faire évoluer le nombre de conseillers communautaires par commune, ça introduit l'idée que c'est forcément par le rapport de force numérique qu'on arrivera à avoir raison et ça, pardon, mais c'est le début de quelque chose qui est sans fin et à ce moment-là, la petite île insulaire qui est rattaché d'interco qui est sur le littoral vont, bref, je pense qu'il faut faire attention à ça, mais j'entends de fait puisque vous avez dit. Merci monsieur le ministre, monsieur Kerrouche. Oui, j'habite également une commune touristique, une commune littorale et a, effectivement, on a répondu partiellement à travers la question du pacte de gouvernance de on a répondu également avec la possibilité de reprise de la compétence touristique pour les stations classées, ce qui fait que, en termes de création de la politique intercommunal, même si j'étais pas d'accord, elles auront plus de latitude, et enfin, il ne faut jamais oublier non plus que l'intercommunalité, toutes choses égales par ailleurs investi beaucoup plus également dans ces communes en matière d'équipements en matière de voirie et donc en gros ça s'équilibre et je je pense pas effectivement qu'aller à l'affrontement numérique suffisent à se faire respecter au sein de l'intercommunalité. monsieur Kerrouche. Chers collègues, souhaitez-vous maintenir vos amendements. Alors, nous allons donc passer au vote sur ces amendements qui ont un avis défavorable de la Commission et du gouvernement qui est pour. Qui est contres. Qui s'abstient ces amendements ne sont pas adoptés, nous passons à l'examen de l'amendement 530 rectifié bis présenté par Madame Noëlle. Merci madame la présidente, monsieur le Ministre, mes chers collègues, le présent amendement a pour objet de rattacher la commune de ces celle dans l'Ain, au département de la Haute-Savoie, comme le ministre ici présent, s'y était engagé auprès de ma collègue Virginie Duby Muller, députée de la Haute-Savoie, lors de l'examen du texte organisant les communes nouvelles et la diversité des territoires, les 2 communes de Seyssel, dans l'Ain et de Seyssel en Haute-Savoie sont géographiquement 1000 limitrophes mais constituent 2 entités distinctes, elles sont situées donc sur 2 départements différents, l'une dans l'un, l'autre en Haute-Savoie, cette modification des limites territoriales des 2 départements concernés est un préalable indispensable à la fusion de ces 2 communes souhaiter à de nombreuses reprises par les 2 conseils municipaux ont voté à l'unanimité de la dernière fois en 2018, les élus de la commune de l'Ain, souhaite rejoindre le département de la Haute-Savoie, qu'il qualifie comme étant leur bassin de vie, ce désir de fusion est le fruit d'un travail commun entre les 2 municipalités qui partagent le même nom, mais qui sont séparés par le Rhône qui matérialise la frontière entre les départements de la Haute-Savoie et de l'Ain, cette fusion permettrait bien sûr d'être plus efficace sur les plans économiques et sociaux de mutualiser les compétences pour maintenir les services publics également bien sûr d'avoir un impact financier positif au-delà de l'identité du nom, clés de communes sont liés par une histoire commune, elle, elle partage de nombreux points, que ce soit au niveau associatif festif, commerciale, artisanale d'échanges commerciaux également de nombreux il existe également des accords inter-départementaux pour la scolarisation des enfants de part et d'autre de la frontière, et enfin il faut noter que le rattachement de la commune du au département de la Haute-Savoie ne portera nullement atteinte à l'intégrité du département de l'Ain, puisque la commune de Seyssel ne représente que 0,0 42 pourcent de la superficie du territoire du département de l'Ain, il en va de même pour la population de ces Seyssel, à savoir 980 un habitant en population municipale au 1er janvier 2017 pour une population municipale de 619497 habitants pour le département, soit 0,15 pourcent seulement de la population du département de l'Ain. Merci, cher collègue Madame la rapporteure, avis de la commission. Merci madame la présidente, de savons traiter ce sujet de création de communes nouvelles à partir de communes situées sur 2 départements différents, nous avons eu un long débat je pense que la proposition qui a été fait par la commission des lois qui va confier à l'État par le biais d'un décret la le règlement de cette décision, né date désaccord de conseils départementaux me permet de dire que votre demande devra être satisfaite et donc c'est une demande de retrait chers collègues. Merci, Monsieur le Ministre. Oui, madame la présidente, on a effectivement discuté avant le dîner, à l'occasion du l'amendement déposé par le sénateur chaises donc effectivement même avis demande de retour. Alors je retirerai mon amendement, l'essentiel étant qu'on puisse sortir de cette situation qui est enlisé depuis de nombreuses années et qui constituent quelque part une forme de tutelle d'une collectivité, sur une autre qui n'est pas acceptable, je remercie. Madame Noël, l'amendement 530 rectifié bis s'est retiré, nous passons à l'examen de l'amendement 768 rectifié, il est présent. C'est

de niveaux d'intercommunalités qui se superposent : la métropole du Grand Paris, puis les OPT s'établissements publics territoriaux qui eux-mêmes sont irrités, pour un certain nombre d'entre eux d'Écossais, des anciens conseillers d'agglomération

où on va flécher là pour le coup, les conseillers métropolitains du Grand Paris, qui sont le plus éloignés des citoyens et on va demander maintenant d'élire les conseillers de péter au sein des conseils et

d'agglomération, pardon, il y avait une réalité existante, donc à ce qu'on demande, je sais que le président de la République va annoncer des choses sur le Grand Paris dans une future énième loi de décentralisation, ce que nous demandons, c'est le gel, parce qu'on ne peut pas demander quelque chose en 2014, avoir un autre type de vote en and dans les échéances qui arrivent, puis après, revenir pour dire on va rechanger encore le système en 2026 nous sommes dans une moment de simplification pour les élus locaux, donc nous demandons le gel, c'est que 11 en flèche, les conseillers territoriaux. Ceux des OPT et que on puisse choisir au sein des conseils et des conseils municipaux, ceux qui iront présenteront donc les conseillers métropolitains, donc c'est un gel, ce que nous demandons, en attendant la grande réforme et l'énième loi de décentralisation qui va concerner le Grand Paris, voilà je vous remercie. Merci beaucoup, madame la présidente, votre présentation est très clairement chers collègues avec le rapporteur nous avons auditionné tous les acteurs de ce que j'appellerai, d'un mot qui n'est pas un mot correspondent à une structure mais le Bassin parisien, nous avons bien compris, je crois que vous l'avez clairement expliqué qu'il y a un certain nombre de difficultés et qu'en tout cas la situation qui a été créé par la loi et très insatisfaisante il y a un accord quasi unanime sur cette situation d'insatisfaction, toutefois il y a pas du tout d'accord sur les solutions à mettre en oeuvre, donc moi j'entends bien ce que vous dites et qu'en même temps il y a pas de consensus aujourd'hui sur ce sujet que nous sommes à quelques mois des prochaines élections municipales, et encore une fois, même si votre proposition est extrêmement justifiée, nous sommes aussi sur un scrutin de Nice il y a une tradition et public and qui consiste à ne pas modifier le mode de scrutin, à quelques mois des élections, donc c'est une demande de retrait ou un avis défavorable et je sais que le gouvernement s'est engagé à à aborder et à traiter cette question extrêmement particulière mais qui n'est pas qu'une situation locale parce que je crois que le sujet que vous évoquez a aussi des conséquences nationales, donc c'est un avis, enfin, une demande de retrait ou un avis défavorable. Monsieur le Ministre, avis du gouvernement. Oui, madame la présidente, on a beaucoup parlé de la loi notre depuis le début de nos travaux, on pourrait aussi effectivement beaucoup revenir sur eux MAPTAM moi ce que je propose, depuis le le début de ce texte, vous le savez, je l'ai dit au sénateur Lafont sénateur Pémezec sénateur Dallier à quelques autres, déjà la semaine dernière, c'est que la question métropolitaine que cela soit d'ailleurs à Marseille, à l'exception près de la question de la voirie, sur lequel il y avait urgence et la question de la métropole du Grand Paris fasse l'objet d'un titre à part entière dans le projet de décentralisation, que l'on va évoquer au 1er semestre de l'année 2020, je suis l'heureux ministre qui a hérité du dossier de la métropole du Grand Paris. Très simple sur lequel je continue les différentes consultations, monsieur le sénateur, tant sur le volet de la gouvernance que sur le volet des compétences et je le crois aussi monsieur le sénateur sur le volet potentiellement du périmètre puisque tout est ouvert, et en tout cas, il y a des propositions dans tous les sens sur l'état du droit, je n'y reviens pas, vous avez rappelé la le double niveau néanmoins les EPT ne sont pas des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, comme la loi commence pas tout ça, on s'en est déjà parlé la semaine dernière donc demande de retrait avec le même engagement que je fais à vous-même, monsieur le sénateur, et à votre groupe, c'est qu'évidemment cette question soit traitée dans le titre global métropolitain que nous serons amenés à à travailler dans la loi de l'année prochaine, je ne souhaite pas ouvrir de brèche les questions métropolitaines sur ce projet de loi puisque au vice au 981 amendement déposé au début de la discussion, nous en reste 365 et si nous avions traité la question métropolitaine, je pense qu'on aurait pu ouvrir la séance, une semaine de plus. Merci monsieur le ministre monsieur Richard, vous avez la parole. Monsieur le président, je suis favorable à l'amendement qui a été déposé par notre collègue et je voudrais faire observer madame la rapporteure, que je me suis exprimé plus d'une fois dans cette maison en commission en séance pour suggérer qu'on ne change pas les règles électorales, la période d'un an et précisément peut-être votre attention a été un peu distraite mais c'est ce que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire que par rapport à l'échéance précédente l'élection dans les intercommunalités existantes en Île-de-France en première couronne se faisait par fléchage, je me permets de solliciter votre attention madame le rapporteur moitié, une grosse moitié comme le disait notre collègue de ceux qui sont devenus les territoires étaient des intercommunalités existantes qui sont devenus les territoires, ils étaient élus par fléchage sur les listes municipales et donc l'application de Le nôtre, aboutit à un changement cette fois-ci, qui franchement n'est pas heureuse,

et on va faire choisir dans les conseils municipaux avec beaucoup moins une garantie de pluralisme les représentants à l'intercommunalité de proximité donc dans l'état d'esprit que le ministre a accepté, à propos de Marseille, c'est-à-dire de ne pas laisser s'engager des situations risque de mal maîtrisée dans un processus métropolitains qui est en cours, je pense que la logique du gel, c'est-à-dire de dire on continue à élire les les intercommunalités de proximité relative, hein, parce que c'est des oeufs intercommunalité de 600000 habitants, mais dans lequel il y aura une certaine pluralité de représentations parce qu'une commune de 50000 habitants et la 5, 6 ou 7 représentants dans le territoire alors qu'un moment à la à à la métropole, donc je trouve qu'il est beaucoup plus cohérent de faire élire par les électeurs, les représentants dans l'intercommunalité, de proximité et de laisser le conseiller choisir 98 90 fois sur 100 le maire comme représentant la métropole, donc je pense que c'est, c'est plutôt une proposition de bon sens.

mais on entend on sera vigilant, on sera dans le débat constructif avec vous, je pense que quand même on pouvait se dire que le fléchage de proximité, c'est-à-dire pour les OPT est quand même une meilleure idée que le fait le fléchage métropolitains qui est quand même une strate au-dessus, voilà, donc là il y a une petite contradiction on aurait aimé, mais j'entends ce que vous nous dites plutôt qu'on aille sur le, sur la même situation que 2014, voilà le statu quo. Parce que là, on avait une situation d'2014 une nouvelle en 2020 et puis sans préjuger des débats que nous aurons entre les à venir des intercommunalités. Ben, on aura certainement une situation nouvelle, en 2026 bon, donc on va, on va le même dire et puis après, advienne ce qu'il adviendra de notre amendement, je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est à Madame Lavarde. Oui merci madame la présidente, alors j'abonde forcément dans le sens de cet amendement, puisque je l'avais déposé en commission des lois commun notre de nos collègues qu'il a été rejeté par la commission et parce qu'effectivement, les établissements publics territoriaux se sont quotidiens, c'est ce que les habitants connaissent, ils ont le logo de l'EPT sur leurs poubelles scellées, le PT qui vient refaire le trou dans la voirie c'est le PT, qui gère les établissements intercommunaux, les conservatoires, les équipements sportifs, la métropole du Grand Paris, elle ne fait rien pour leur quotidien, si vous demandez la main Francilien, ce qui connaît la métropole du Grand Paris, j'en suis pas sûr parce que ce n'est pas son son organe de proximité, je vais vous donner un exemple dans ma ville, nous avons 21 conseillers territoriaux donc qui seront désignés demain par le conseil municipal plupart fléchage donc les les citoyens ne pourront pas s'exprimer sur les gens qu'ils envoient, nous avons 3 conseillers métropolitains, donc vous voyez bien que les proportions sont absolument pas les mêmes donc enfin effectivement et en plus on ne change pas les règles du jeu à à 6 mois Merci, la parole est à Madame Gatel. ce que j'ai voulu dire aujourd'hui c'est que on ne change pas les règles, à quelques mois des élections parce que la règle que vous demander de geler, elle n'a certes pas été appliqué aux élections de 2014 puisqu'elle est postérieure à ces élections, mais c'est la loi, notre. Qu'il a fixée, donc ça veut dire que la loi a après l'élection de 2014 mais bien avant celle de 2020 défini les conditions d'élections sur lesquelles vous émettez et j'entends parce on a entendu ces expressions un grand nombre de réserves, donc ce n'est pas ce que la commission propose ce soir qui vient changer les règles, la commission dit que, à quelques mois des élections au nom de cette tradition républicaine en plus sur un scrutin de listes il nous sommes extrêmement difficile de changer une règle qui sans doute est justifié mais qui ne fait pas consensus, donc voilà, je tenais à ce que le message soit clair, chers collègues, je craignais de mètres fait mal comprendre. Merci madame la rapporteure monsieur Roger a demandé la parole. Oui, rapidement pour dire que, comme les autres collègues, Alain Richard, Fabien je suis tout à fait à penser qu'il vaut mieux, dans une grande sagesse laisser nos électeurs qui sont déjà perdus sur le lien commune pt moi je suis d'Est Ensemble c'est 450000 habitants, donc c'est déjà compliqué à comprendre alors le Grand Paris, ils savent pas du tout ce que c'est et donc la sagesse serait de ne rien toucher et d'attendre le débat qui était annoncé par le ministre et qui va nous permettent peut-être d'essayer de trouver une solution commune dans ce grand bassin parisien voilà. monsieur Roger s'il n'y a plus de demandes de prises de parole, je vais mettre aux voix cet amendement 768 rectifié qui, avec une demande de retrait de la Commission et du gouvernement qui est pour. Qui contrent. Qui s'abstient l'amendement n'est pas adopté, nous passons maintenant à la présentation. De. 8 amendements qui font l'objet d'une discussion commune le 1er présenté par Madame Berthe et. Oui, je vous remercie, madame la présidente, madame et monsieur le rapporteur, monsieur le ministre, mon amendement vise, j'allais dire, simplement mais à réduire le nombre d'élus locaux dans les communes afin de faciliter la constitution de listes pour les élections municipales, il est motivé par les retours d'une grande partie des élus de mon département de la Savoie, petite ou grande commune, quelle que soit leur taille. Merci madame Woerth et nous passons maintenant à monsieur Pacaud qui va nous présenter le 327 rectifié terre. Merci madame la présidente, monsieur le ministre, chacun sait combien il est compliqué de composer des listes de personnes motivées, impliqués dans la vie des communes de petite taille, certains acceptent de s'y inscrire, pour faire plaisir, pour boucher les trous, mais une fois élu, viennent rarement et même parfois plus du tout le présent amendement vise à assouplir les règles numérique strictes pour la composition de liste à l'occasion des élections municipales assouplir, et non pas réduire la plupart des autres amendements visent à une réduction obligatoire, moi je préfère la souplesse et la possibilité de réduction, mais la possibilité aussi de maintien au stade actuel, la possibilité, dans l'obligation de réduire légèrement le nombre d'élus sans affaiblir sensiblement la possibilité d'éligibilité des citoyens des communes de petite taille et sans affaiblir l'efficacité de l'équipe municipale doit pouvoir faciliter la qu'on alors concrètement, qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que dans une commune de moins de 100 habitants, je propose des conseils de 9 ou 7 personnes dans des communes de 100 à 499 habitants 9 ou 11 personnes et ainsi de suite, on on remonte jusqu'aux communes de 3500 à 4999 habitants où on aurait des conseils de 25 ou ou 27, alors vous allez me dire, mais entre les 2 chiffres, lequel va-t-on choisir, hé bien il y a un alinéa dans mon amendement qui le précise le nombre définitif des membres du conseil municipal et le nombre maximal prévu sauf si aucune liste ne présente autant de candidats dans ce cas, c'est le nombre minimal qui sert de référence concrètement un exemple, une commune de 1100 habitants, vous avez 2 listes de 13 membres qui se présente, vous aurez un conseil de 13 membres, vous avez une liste de 13, une liste de 15 vous aurez un conseil de 15, voilà le but c'est vraiment d'assouplir. éventuellement de réduire ce qui peut permettent de faciliter la constitution de certaines listes, mais de ne pas rejeter toutes les bonnes volontés, quand vous êtes capable de remplir, entre guillemets, votre liste sans aucune difficulté, que vous avez toutes les bonnes volontés pour il faut les garder Merci monsieur Pacaud, la parole est à madame vu lien pour le 501 rectifié bis. d'amendements qui, qui concerne aussi cette crise des vocations qui est constatée dans de nombreuses communes, notamment des communes de petite taille, alors ce que nous proposons, nous, c'est un petit peu différent, donc il faudra choisir un moment donné, c'est pour faire enfin cette situation, l'objet de cet amendement vise à baisser le nombre de conseillers municipaux de 7 à 5 pour les communes de moins de 100 habitants de 15 à 13 dans les communes de 500 à 1000 400 99 et de 19 à 17 dans les communes de 1500 à 2499 ce qui permettrait sans doute de trouver plus facilement des citoyens qui veulent s'engager pour leur commune, je vous remercie. cet amendement vient en écho à un amendement antérieure que j'ai proposée qui permettait des listes proportionnelles et qui demande à ce que les listes soient proportionnels à partir de 200 habitants un écho à ceux-là, pour que des listes puissent se constituer, j'ai proposé et c'est l'objet de cet amendement, un abaissement du nombre de conseillers par liste, ce qui favoriserait et la parité pour les le fait que les listes soient proportionnels, mais aussi la capacité à former des listes, voire d'autres listes, puisqu'on a remarqué que le fait de mettre des listes à la proportionnelle, à partir de 1000 habitants, con comme considérablement la capacité à faire des listes concurrentes dont moi je propose un abaissement des élite pour pouvoir justement faire et qu'il y ait plus de démocratie. Merci monsieur Marc nous passons 579 rectifié bis, il est présenté par Monsieur Lluch. Oui, madame la présidente, monsieur le le ministre mais mesdames et messieurs les rapporteurs, cet amendement vise à son tour à augmenter le seuil de 100 à 200 habitants pour obtenir des conseils municipaux, 7 membres, il existe un effet, ça a été rappelé de réelles difficultés, constitué de ces conseils municipaux dans des très petites communes par exemple ce pot nous commune samedi habitants juste le cap des 100 habitants au-dessus, trouver des personnes pour réaliser une caution municipale de 11 membres, relève d'une mission purement délicate cet cet amendement propose de faciliter la vie des telle petite commune avec quoi ça municipal réduit et qui sera plus facilement opérant. Merci monsieur Luche, maintenant nous passons 804 rectifié bis et c'est madame Cukierman qu'il présente. Merci madame la présidente, monsieur Miss cet amendement va peut-être un peu à l'encontre des précédents et pour autant, il s'appuie aussi sur des réalités, puisque je crois dans la discussion, en tout cas avec un certain nombre de maires de communes de moins de sens habitant ils font apparaître aujourd'hui la difficulté à avoir effectivement le nombre de conseillers municipaux, réduit à 7 pour plusieurs raisons : d'abord parce que il y a des effets au bout d'un mandat qui sont inhérents finalement quel que soit le nombre de conseillers municipaux, au fait que, il y a toujours une ou 2 personnes qui peuvent être amenés à changer de vie a changé de lieu de vie et donc, bien évidemment, quand on commence à 9 et confiné à 7 c'est toujours plus facile quand on commence à 7 et qu'on finit à 5 et que l'on le, on le sait, c'est justement dans ces plus petites communes que l'importance que l'ensemble des conseillers municipaux et de leurs nombres puissent être présents tout au long, tout au long du mandat pour ne pas faire peser une fine et à la fin des 6 ans sur un, 2 ou 3 élus dans les faits, la gestion des affaires communales, donc c'est pour cela que nous proposons finalement de revenir à ce qui existait antérieurement à savoir pour les communes de moins de 100 habitants le passage de 7 à 9 conseillers municipaux. Merci madame la présidente, à travers l'ensemble de ces amendements sont que confusément, il y a une difficulté avec la représentation dans les communes de moins de 1500 habitants et un questionnement autour donc du nombre de de conseillers qui serait utile à en tout cas, complètement impliqué, on va dire dans la vie, dans la vie locale, pour notre part, nous considérons que la strate des communes entre 500 et 1499 habitants qui rassemble 28 pourcent des communes françaises rassemblés communes qui ont des profils malgré tout très différents et elles sont traités de manière identique et nous proposons donc un barème plus progressif avec une strate entre 500 et 999 habitants et une autre de 1000 à 1499 habitants toujours dans la perspective d'une progression plus moins rapide du barème et de la possibilité de trouver donc assez de conseillers municipaux.

Merci madame la présidente, monsieur le ministre, c'était amendement est une réponse aux inquiétudes des maires des communes de moins de 500 habitants qui craignent un nombre insuffisant de candidatures pour le prochain renouvellement et qui craignent de ne pouvoir satisfaire le le nombre de conseillers municipaux, une nouvelle refonte des seuils n'a pas été envisagée ici comme ça a pu être présenté dans les amendements précédents parce qu'une refonte des seuils produiraient des effets similaires, tant en Avantage qu'on inconvénient : ce qui vous est proposé, c'est un système dérogatoire en permettant que les conseils municipaux des communes de moins de 500 habitants soit réputés complet au terme d'un scrutin municipal qui n'aurait pas désigner un nombre suffisant de conseillers municipaux, sans que ce nombre ne puissent être inférieure à 5 conseillers municipaux dans les communes de moins de 100 habitants est inférieur à 9 conseillers pour les communes de 100 à 499 habitants cet amendement apporte une nuance au logique de seuil sans pour autant pénaliser les communes qui aurait la capacité de réunir suffisamment de candidatures et donc d'élus, je vous remercie. Merci. Alors merci, cher collègue, maintenant nous passons à la présentation par monsieur le ministre du sous-amendement donc numéro 980. merci madame la présidente, peut-être aurions-nous dû avec la commission, faire une prise de parole préalable sur l'ensemble de la discussion commune de de ces amendements. 16000 communes ont moins de 500 habitants donc ce que nous allons faire mérite comme sa plus grande des attentions, puisque ce n'est pas neutre de est ce que l'on doit avancer avec plus de souplesse pour permettre justement cet engagement, la réponse est oui, 3, la vraie question au travers cette discussion commune, on le voit bien, c'est le caractère réversible ou irréversible de ce que nous faisons si vous diminuez définitivement le nombre de conseillers municipaux sur une catégorie ne reviendront pas en arrière et on sait très bien aussi que, dans certaines communes il y avait pas de problème pour compléter le conseil municipal dans cette commune, vous avez un problème sur une série de type 2020, vous pouvez avoir des difficultés à boucler la liste, puis la série 2026 vous pouvez de nouveau avoir des candidatures, sauf qu'il se trouve que le moment vous avez sorti votre tuteur pour commencer à. Diminuer le nombre de, de, de postes de conseillers municipaux dans un conseil municipal, une fois que vous avez commencé le régions vous avez commencé à le réduire, c'est pour ça que quand j'ai vu et lorsque nous avons examiné l'ensemble des amendements en lien avec la commission des lois telles que vous ne les avait présentés mesdames messieurs et sénateur, le sénateur de madame l'amendement de la sénatrice de Seine, pardonnez-moi, c'est triste, est un amendement intéressant parce qu'il tient compte de cette, de ce caractère réversible de la mesure et donc en clair ce que nous proposons, par ce sous-amendement pour venir le compléter avec votre permission, mais à la sénatrice de venir dire au fond. Lorsqu'un conseil municipal n'est pas réputé complet aujourd'hui, vous avez un certain nombre de d'actes qui ne sont pas possibles, et non des moindres, notamment l'élection du maire, ce qui déclenche donc des partielles, parfois à tout moment, même pendant le mandat, y compris d'ailleurs parfois plusieurs fois dans la même commune pendant le mandat ou en tout cas, même parfois quelques semaines avant le renouvellement général et donc l'expérience l'expérimentation que je vous propose par ce sous-amendement en s'inspirant et en s'appuyant sur votre amendement madame la sénatrice c'est permettre de faire que pour les communes de moins de 500 habitants lorsque le Conseil n'est pas complet, on leur est plus complet, ce qui est donc et réversible évite de supprimer un certain nombre de postes de conseillers municipaux fait que bah le Conseil fonctionne avec ce que la collectivité locale, avec ce que le territoire en question a trouvé comme comme la 2ème des choses que je propose dans le sous-amendement, c'est de garantir un minimum de conseillers municipaux, pour des raisons éminemment constitutionnelle 4 à 5 conseillers municipaux 5 la durée du la durée du mandat quatre la dernière année du mandat, ce qui correspond à la situation telle qu'on peut la connaître parfois aujourd'hui, et là vous avez un dispositif qui robuste, il faudra voir comment il vit, il me semble, pragmatique et elle permet de répondre à mon avis aux aspirations et aux attentes du Sénat sur les différents amendements que vous avez que Dernier point, je ne suis pas certain qu'il y a un consensus aussi large que cela. à diminuer le nombre de conseillers municipaux dans les communes rurales dans notre pays, on le pose comme ça, nuitamment, je l'avais indiqué en discussion générale si véritablement il y avait un accord politique de tous les groupes politiques ici au Sénat le gouvernement était à la disposition du Sénat pour regarder cette affaire de près, mais enfin des débats que nous avons pu avoir déjà depuis maintenant plus de 10 jours, je vois bien que non, et donc la solution, s'appuyant sur l'opportunité de votre un moment mais elle va sénatrice à mon avis est une solution de compromis qui me semblent intéressantes et qui permettra, à mon avis de suppléer aux difficultés d'engagement que l'on peut avoir sporadiquement dans telle ou telle commune rurale en tout cas je pense que l'amendement ainsi sous-amendé est donc une oeuvre de bon sens. Et monsieur le ministre, la parole est à madame le rapporteur pour la vie de la commission. des questions et des enjeux, et notamment l'amendement 44 et le sous-amendement puisqu'en présentant son sous-amendement, monsieur le ministre, a présenté l'ensemble du sujet qui consiste à traiter la question compliquée de l'effectif d'un conseil municipal sur lequel il a dit à ce stade, il n'y a pas de consensus des associations mais il nous faut traiter la question difficile et délicate de certains conseils aux municipaux réputé incomplet. Donc là, les amendements, alors je vais les prendre dans l'ordre si vous voulez bien, donc les amendements 659 rectifié bis 327 rectifié terre 501 rectifié 648 rectifié 570 neuf rectifier bis et 400 rectifié bis tendent tous à modifier la composition des conseils municipaux pour diminuer le nombre de conseillers dans les petites communes sous des modalités différentes, la commission il est défavorable pour différentes de région, on n'est pas certain d'abord que la crise des vocations que traversent certaines communes qui ont du mal à disposer d'un nombre suffisant de conseillers municipaux choix permanente, il n'est donc pas exclu que des communes rencontrant ce type de difficultés et parfois un nombre suffisant de candidats en tout cas, tout cela doit nous inciter à une grande à une deuxièmement, il semble que la solution qui consiste à le conseil communal complet, même s'il ne dispose pas de tous ses membres, pourrait apporter une souplesse aux communes en difficulté sans pénaliser les autres et c'est cette idée de solutionner les cas difficiles, sans créer d'impact négatif sur les autres Par rapport aux autres amendements que j'ai évoqué l'amendement 44 de notre collègue de seuil, nous sommes comme au gouvernement, un amendement extrêmement intéressant, sachant qu'il y a une proposition du sous-amendement par le ministre sous-amendement auquel la Commission est favorable,

600 48 et 579 qui ne sont pas compatibles amendement proposé par notre collègue de et pour les autres, donc 327 et 401 ce sera également un avis défavorable car il pose d'autres questions et sur l'amendement 800 cas de rectifier bis qui lui tend à relever le nombre de conseillers municipaux dans les communes de cette de 100 habitants de de moins il pourrait créer un certain nombre de difficultés dans certaines communes, donc c'est un retrait ou à défaut un avis défavorable à l'amendement 800 cas j'espère avoir été. Pierre Mazars rapporteur interne Monsieur le ministre pour l'avis du gouvernement. Oui, madame la présidente, je t'encore plus bref avis défavorable aux demandes de retrait pour l'ensemble des amendements, sauf le 44 rectifié, terre de madame de scène avec le sous-amendement présenté par le gouvernement. Merci monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des lois, vous avez la parole. Madame la présidente, je demande la priorité de vote sur l'amendement numéro 44 rectifié, terre de Madame de Seine, ainsi que sur le sous-amendement du Gouvernement numéro 980 1 à cet amendement. Merci. Si Monsieur le Président, je suis donc saisie d'une demande de priorité de la commission sur l'amendement numéro 44. Pour rectifier terre et le sous-amendement 981 tendant à insérer un article additionnel après l'article 11 qu'inquiet s'afin qu'il soit mis aux voix en 1er selon l'article 44 à Lille est née à 6 de notre règlement. La priorité est de droit quand elle est demandée par la commission, saisie au fond, sauf opposition du gouvernement, quel est donc l'avis du gouvernement sur cette demande de priorité Monsieur le Ministre. Quel suspense, la vie est naturellement favorable. Alors, la priorité est ordonnée, je vais donc mettent. Anne Sicile. Je mets aux voix maintenant le sous-amendement 980 Explications de vote de Madame Cukierman. Je vous remercie, madame la présidente, monsieur unissent, mes chers collègues, c'est une explication de vote qui viendra pour le sous-amendement et l'amendement qui effectivement sont certainement une solution de compromis, nous allons voter cependant à Madame la rapporteure, n'y voyez aucune malice, mais nous nous adaptons nous faisons évoluer, nous permettant de la souplesse, à quelques mois des élections municipales, alors que le scrutin était clairement définie pour les communes identifiées, donc je voudrais pas qu'il est, donne entre des des établissements des groupements d'Île-de-France et et des communes rurales, donc je voudrais qu'on puisse repréciser très précisément ce qu'il en est, pour ne pas donner le sentiment que sur certains amendements, il y aura un avis défavorable ou de retrait parce que nous serions à l'approche d'une séquence électorale et que pour d'autres cela ne poserait pas de problème, je vous remercie. Merci madame Cukierman il n'y a pas d'autres demandes. Et explications de vote de Monsieur Queiroz. Oui, nous sommes que les 2 l'amendement et le sous-amendement présente une solution intelligente que nous voterons. Merci, alors Madame Catala, demandé la parole sous-amendé par le gouvernement n'est pas une modification du mode de scrutin, contrairement à ce que nous avons abordé tout à l'heure au sujet du de la métropole et des ETP. Merci madame guêtre celle. Il n'y a plus de demandes d'explications de vote, je vais donc mettre aux voix le sous-amendement 980 qui est pour.

Quiconque. S'abstient, il est adopté. Nous avons un donc un amendement 659 rectifié bis qui tombe.

Bien entendu les arguments de Madame le rapporteur, simplement, j'étais un petit peu gêné d'entente que cet amendement le 327 prévoyait, comme les autres, une réduction du nombre de

Qui est contre. Qui s'abstient, il n'est pas adopté le 100 101 rectifié bis tombe le 648 rectifié tombe

Qui est contre. S'abstient, il n'est pas adopté et enfin je mets aux voix le 401 rectifié bis qui est pour. Qui est contre. Qui ça, il n'est pas adopté, nous passons à l'examen de 2 amendements. Identiques faisant l'objet d'une discussion commune et nous commençons par le 400 rectifier bis présenté par monsieur Monsieur Durand. Ce sera bien aussi, madame la présidente, notre collègue Kerrouche est allé chercher puisée aux meilleures travaux du du Sénat puisque c'est dans une proposition de loi relative à l'équipe territoriale et à la vitalité de la démocratie locale, déposée par messieurs bah Retailleau d'Arnaud et dans son article 21 ter que nous trouverons une solution une difficulté qui est souvent rencontré dans les conseils municipaux, puisque comme le dit Woody Allen l'éternité, c'est long. Surtout vers la fin et les mandats municipaux sont parfois, eux aussi, très très long, surtout vers la fin, puisque quand conseiller municipal vient à faire défaut à démissionner et qu'il s'agit donc d'une incomplétude du conseil municipal et qu'il faut remplacer le maire ou un adjoint, il n'y a pas d'autre solution que de procéder à une élection municipale partielle à une Renault un renouvellement dans son intégralité du conseil municipal, municipal, donc la solution qui est proposé, c'est qu'on puisse proposer pour procéder à l'élection du maire, en dépit de la complétude du conseil municipal jusqu'à 10 pourcent de ses membres. Merci, merci beaucoup, Monsieur Durand. Monsieur chaises va présenter son amendement. Oui, madame la présidente, monsieur le ministre, en fait, cette exactement le même amendement j'allais dire que c'est l'expérience malheureuse d'une élection qui s'est passé après une démission du au cumul des mandats, qui m'a fait donc rédigé cet amendement en fait à l'élection de 2014, une seule liste étaient présentes donc en lice dans la commune si veux dire qu'il n'y avait aucun remplaçant par malheur un des conseiller municipal est décédé ce qui fait que, au moment de l'élection du maire, il a fallu refaire des élections complète, outre le fait que évidemment c'était événement et complexe, elle est aussi assez traumatisante pour les élus qui a été élu pour un mandat de 6 ans et qui ont dû s'arrêter brutalement au bout de 4 ans de part gérer un artifice électoral.

parce qu'ils permettent de gérer les situations doit élire un maire alors le constat : alors que le conseil municipal est incomplet, sachant que l'incomplétude et de l'ordre de 10 pourcent de de ciment, donc c'est un avis favorable. Merci madame la rapporteure, Monsieur le Ministre. Oui, madame la présidente, alors tout le monde s'inspirer et donc tout le monde puisse dans les meilleurs travaux tout le monde et je m'en réjouis, une forme d'économie circulaire, une forme de de mise en consigne des rapports sénatoriaux et restitution à leurs auteurs, la suite des amendements qui feront l'objet d'une discussion commune me semblait peut-être par la rédaction plus plus plus opportune sagesse à vrai dire, sur sur ces amendements et je ferai un avis favorable sur l'ensemble des amendements qui suivent. Merci monsieur le ministre madame Guillemot a demandé la parole pour explication de vote ah bon. Nous allons passer au voit donc sur ces amendements qui ont un avis favorable de la commission et un avis de sa chaise du gouvernement qui est pour. Qui contrôle. Qui s'abstient ils sont adoptés. Nous passons maintenant à l'examen de si les amendements faisant l'objet d'une discussion commune le 1er le 8 rectifié, sexe, yes et présenté par Monsieur Madame la présidente, monsieur, lui, je vais faire, collègues, il s'agit par cet amendement de permettre, en cas de décès ou démission d'un maire de procéder à une nouvelle élection avec une liste incomplète ou un conseil incomplet ceci pourra se faire à à moins de 18 mois du prochain renouvellement l'article L 21 22 8 prévoit que pour l'élection du maire, le conseil municipal doit être complet et que si une telle n'était pas le cas, il doit être organisé des élections complémentaires afin de mettre fin à la vacance des sièges, il est souvent compliqué de le faire dans les petites communes, cet amendement tend à répondre à une demande forte des maires des communes, notamment rurales qui sentent lorsque le Conseil a subi des défections c'est un donc un un demande de simplification, limité à 18 mois avant les élections. la parole est à monsieur Kern, pour présenter le 53 rue. Six fiottes. Merci madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, j'ai le plaisir de défendre cet amendement de mon collègue Vincent Delahaye est à l'initiative, il vise à remédier à une situation que de nombreuses communes rencontrent, à savoir l'obligation d'organiser une élection municipale, suite au décès ou à la démission du maire, quand bien même cela interviendrait moins d'un an avant l'organisation des élections municipales générales dans le département de l'Essonne, telle fut récemment le cas à Verrières-le-Buisson, suite au décès de son précédent maire en effet la loi dispose que le conseil municipal doit être complet afin de procéder à l'élection du maire et ce à tout moment du déroulé du monde ainsi les communes dans lesquelles le maire n'est plus en mesure d'occuper ses fonctions peuvent être tenus d'organiser des élections municipales partielles, très peu de temps avant les élections municipales générales. Or de telles élections représentent un coût non négligeable pour les communes, par ailleurs, eu égard à l'importante proximité temporelle entre l'élection partielle et l'élection générale, les électeurs peuvent ressentir moins d'intérêt pour le scrutin, cet amendement entend remédier à ces inconvénients, réservant l'obligation d'organiser des élections municipales partielles dans l'année précédant les élections générales afin de procéder à l'élection du maire au seul cas où le conseil municipal aurait perdu plus d'un tiers de ses membres. Si Monsieur Kern, nous passons à l'examen de l'amendement 380 rectifié monsieur de Belenet.

Oui, madame la présidente j'explique d'abord pourquoi j'ai été amené un 1er a déposé un amendement que j'ai ensuite rectifié par 2 fois, tout récemment, dans mon département de l'Aude, le maire d'une toute petite commune, celle de Niort, de sauts est décédé, il doit donc être procédé à l'élection de nouveau maire, dès lors, la préfecture demande département à l'application de l'article L 21 22 tiré 8 du code général des collectivités territoriales, indique qu'il doit être procédé avant l'élection du maire à une élection partielle afin de compléter le conseil municipal, or, comme chacun le sait, les élections municipales auront lieu dans environ, c'est moi, il m'est apparu absurde que l'on procède à des élections partielles quelques mois juste avant le renouvellement général, d'où l'amendement que j'ai souhaité déposé avec le soutien du groupe socialiste le droit actuel ne prévoit que de dérogations à ce principe, l'élection du maire peut ainsi se tenir malgré un conseil municipal est incomplet si les vacances suivent immédiatement le renouvellement intégral du conseil municipal d'une commune de 1000 habitants et plus, ou si, à la suite de l'élection complémentaire de nouvelles vacances se produisent et, dans ce dernier cas, le conseil municipal doit conserver plus de 2 tiers de son effectif, il n'existe actuellement aucune règle, évitant de convoquer une élection partielle rendue nécessaire par l'élection du maire à l'approche des élections municipales, ainsi des élections partielles peuvent peut-être être convoqué à quelques mois voire quelques semaines du renouvellement général et cette situation coûteuse pour les derniers, les deniers publics est incomprise par les citoyens qui doivent se déplacer aux urnes à intervalles rapprochés alors que pour l'élection partielle un seul siège peut-être à pourvoir la maintenant initial que j'avais déposé ce proposés dans d'assouplir l'obligation d'un effectif complet du du conseil municipal dans l'année précédant le scrutin, c'est-à-dire le 1er mars, j'avais noté d'ailleurs que ma préoccupation était largement partagée par plusieurs groupes parlementaires, cela dit, il convenait d'élargir cet assouplissement à l'ensemble des communes, sauf évidemment si le conseil municipal a perdu plus du tiers de ses membres, ce fut l'objet

madame la rapporteure, chers collègues, c'est dans le même esprit, on est tous confrontés dans nos départements, à des situations absolument incroyables, ça se passait le week-end dernier, effectivement, le maire est décédé, première adjointe est décédé, à quelques mois de de du renouvellement, on doit ré-élire l'ensemble de l'équipe municipale au-delà du, du coup, c'est plutôt l'incompréhension et quelque part l'irrespect vis-à-vis des de l'équipe municipale pendant qu'il a fait son travail pendant 5 ans, on est à la veille du renouvellement et je trouve qu'il est quand même et fils qui était effectivement très difficile d'admettre que cette équipe qui a parfois d'ailleurs dans beaucoup de cas suppléer l'absence du maire parce que dans les les cas qu'on connaît tous, c'est souvent pour maladie et je trouve que c'est assez irrespectueux, d'où cette proposition de dire qu'on ne renouvelle pas le équipe du conseil municipal l'année précédente, au 1er janvier précédente aller aux élections, de manière à reconnaître le travail qui a été effectué dès lors que les le nombre de conseillère de conseillers ne dépasse pas le tiers des membres, je présente peut-être le suivant, tout à fait le suivant, c'est un amendement de repli, parce que le 1er ces absences du maire qui pourrait provenir d'une démission

le 2ème amendement c'est un amendement de repli qui ne prend en considération, effectivement, que les décès où là effectivement on peut pas être en situation de crise ou de conflits à l'intérieur de l'équipe municipale, donc c'est un tas d'amendements de repli.

donc les amendements 484 8 380 930 et 53 tendent à prévoir une dérogation à l'obligation de convoquer des élections partielles l'année précédente, celle du renouvellement général lorsqu'une vacance de sièges empêche d'élire un ces amendements semble pour nous relever du bon sens et contribuerait, comme cela a été dit par notre collègue Rémi à rendre plus lisible la vie politique locale en tout cas moins incompréhensible pour nos concitoyens, en effet, les appelés aux urnes à 2 reprises à quelques mois d'intervalle ne répond à aucune nécessité politique et perturbe vraiment nos concitoyens, ils tendent également à préciser, lorsque c'est applicable et je vous épargne la liste le seuil de déclenchement d'une élection partielle lorsque l'assemblée délibérante en question a perdu la moitié ou plus, ou bien le tiers au plus parce qu'on respecte ses quotas de ses membres, selon les cas, donc il précise, lorsque c'est applicable, là où les nouvelles éviction sont obligatoires, donc là aussi cette clarification apporte une harmonisation plutôt bienvenue des rédactions au sein du code électoral, ces amendements ayant été rendu identique, ils apportent de la souplesse dont on a besoin pour des situations extrêmement particulière et améliore en même temps la sécurité juridique des collectivités, ce qui n'est pas négligeable à prendre en considération, donc c'est un avis favorable à l'ensemble de ces amendements, donc j'aurai pas 424 8 380 939127 et 53 en ce qui concerne l'amendement 927 mon cher collègue Gremillet, je partage tout à fait votre intention d'attirer notre attention sur le cas spécifique du décès des mères qui crée une situation tout à fait particulière qu'il faut prendre, donc on est sur le plan juridique, il est satisfait, donc c'est une demande de de de retrait que je formulerai Monsieur Guérini. Monsieur le ministre à vie du gouvernement. Oui, madame la présidente, comme je disais tout à l'heure : avis favorable pour l'ensemble des amendements et évidemment demande de retrait pour le le 927 de monsieur Grenier, puisque si le le Sénat adopte l'amendement précédent il sera satisfait.

Oui, je voudrais simplement soumettre à votre sagacité le cas suivant nous avons puisque vous avez refusé d'avoir des listes à la proportionnelle, jusqu'à 200 nous avons le cas suivant une liste à à 8 candidats qui ont été élus, la liste Beane 7 et le maire qui est élu, bien sûr, à la tête de la liste, a malheureusement meurent, nous nous trouvons 7 à 7 nous nous trouvons à un an des élections, donc il n'y a plus d'élection

qui va être élu pour ce qui confère à la liste qui a été battu, un Avantage considérable en attendant les élections à venir, donc moi je proposerai peut-être quelque chose qui serait ça c'est des cas auquel on n'a pas pensé jusqu'à présent, et nous on y a pensé, parce que nous aussi, nous allons nous sommes trouvés dans ce cas-là en Aveyron il y a peu, peut-être vaudrait-il mieux que le premier adjoint ou le second si le 1er malheureusement décèdent aussi assumer les fonctions de maire jusqu'aux élections, plutôt que de procéder à une élection pour devenir pour pour pour élire le nouveau maire, parce que ça peut poser des problèmes puisqu'on peut se retrouver avec l'inverse de ce qu'avait souhaité les électeurs en première intention. Merci, merci, cher collègue, s'il n'y a pas de demandes de parole je vais mettre aux voix. Les 5 amendements identiques qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient ces cinq amendements sont adoptés. Monsieur Gremillet concerne il tombeau et de. Non, non, mais il est flagrant je j'avais pris la précaution de le dire, c'est un amendement de repli dès lors qu'il est satisfait enfin très bien. Ensuite, nous passons à l'examen du 391 rectifié, il est présenté par Monsieur Oui, madame la présidente, il s'agit d'un article additionnel qui serait ainsi rédigé au moins une fois par an, le chef de la circonscription de sécurité publique présente devant le conseil municipal de chaque commune de sa circonscription, l'action de l'État en matière de sécurité et de prévention de la délinquance pour la commune concernée cette présentation est suivie d'un débat, vous le savez, la sécurité est quelque chose de partagé entre les services de l'État, police ou gendarmerie selon les circonscriptions et les collectivités territoriales qui participent et finance, je sais qu'il nous a dit aussi qu'il y a des conseils de prévention de la délinquance, ça n'est pas dans toutes les communes, ça fonctionne entre professionnels de façon discrète et en tout cas ça ne permet pas à la pluralité des conseils municipaux de savoir comment l'État travaille en bonne symbiose avec les collectivités dans le domaine de la sécurité, voilà, j'ai essayé de résumer, pour être court. Merci monsieur Roger, monsieur le rapporteur, vous avez la parole pour l'avis de la commission. Oui, madame la présidente, c'est une idée qui nous est apparue comme une idée particulièrement intéressante, considérant qu'en dehors des c'est il y avait parfois la nécessité de s'adresser directement aux élus municipaux sur des sujets qui les concernent au 1er chef et ce sera donc un avis favorable. Merci, monsieur le rapporteur, monsieur le Ministre. Oui, mais à la prison son avis de sagesse. Merci bien je mets donc aux voix le 391 rectifié avec un avis favorable de la commission et ça Jésus gouvernement qui est pour. Qui et contre qui. S'abstient l'amendement 391 rectifié est adopté le 574 rectifié bis et présenté par Monsieur Leroy. Oui, madame la présidente, monsieur le Ministre, mes chers collègues, ma sécurité, effectivement, ne cesse d'augmenter dans notre pays, c'est bien sûr et d'abord de la responsabilité de l'État, qui dispose du concours des forces de sécurité intérieure pour faire respecter l'ordre mais les maires ont également un important rôle à jouer en la matière il coopère avec les autorités nationales, ils ont la qualité d'officier de plus judiciaire et en le concours de la police municipale, même s'ils ont pas d'habilitation du procureur de la République et de circonscription d'action judiciaire l'article L 22 11 tirer un du Code général des collectivités territoriales, précise que le maire concourent à la politique de prévention de la délinquance, l'amendement que je propose, a pour objet de préciser dès cet article du code que le maire est aussi officier de police judiciaire alors les maires sont en première ligne pour combattre les incivilités, la sécurité, cette précision me paraît utile et nécessaire, merci. Oui, mais à présent je comprends tout à fait des motivations de notre collègue Henri Leroy pour autant le statut d'OPJ et du maire et 2 de ses adjoints et déjà fixé par la loi à l'article 16 du code de procédure pénale sera donc une demande de retrait ou à défaut un avis défavorable. Merci, monsieur le rapporteur, monsieur le Ministre. Même avis mais la présidente. Très bien monsieur le roi vous souhaiter maintenir votre amendement, vous le retirer. L'amendement 574 est retiré, nous passons à l'examen de 2 amendements faisant l'objet d'une discussion commune le 723 rectifié présenté par madame Guillemot pour commencer. Merci madame la présidente, monsieur le Ministre, mes chers collègues, l'amendement le 1er donc, le 723 rectifié a déjà été voté à l'unanimité, à l'unanimité lors des débats sur la PPL visant à améliorer la lutte contre l'habitat insalubre et dangereux, adoptée au Sénat, que nous avons tous à l'unanimité, je le rappelle, le 11 juin 2019, c'est pour ça que je suis assez surprise de l'avis défavorable de la commission des lois, qui vient de nous donner donc cet avis défavorable, je rappelle que nous souhaitions donner de nouveaux pouvoirs aux élus et aux maires qui sont en premières lignes pour lutter conte l'habitat indigne, cet amendement permet aux maires d'intervenir en urgence pendant la période d'instruction du dossier pour préserver la santé ou la sécurité des occupants jusqu'à la prise d'un arrêté de police administrative spéciale qui suppose en pratique un certain délai de 6 mois, 9 mois phase contradictoire réelle réalisation d'échange : nomination d'un expert etc lorsque l'instruction d'un dossier pour logements indignes est enclenché, quelle que soit sa nature péril coin propos insalubrité, le maire doit avoir la possibilité de prendre des et c'est pour ça que nous étions unanimes, vu la situation, qu'il y a aujourd'hui dans notre pays en fonction des circonstances, parce que c'est lui qui connaît le mieux, il est bien évident qu'il va prendre un arrêté s'il pense qu'il ne faut pas prendre cet arrêté et donc toute mesure conservatoire pour protéger au besoin les occupants, il pourrait donc utiliser ses pouvoirs de police générale pour ordonner le relogement et surtout ce qui nous importait c'est la suspension du paiement des loyers, parce que je rappelle que quand le maire prend un arrêté, ça dure 6 mois, un an, hé bien les gens, même s'ils ont un péril parce qu'il est pas imminents, il continue à payer le loyer et nous pensions tous que dans ce cadre-là d'instruction du dossier et bien sûr en faisant confiance au maire, il ne fallait pas laisser les familles dans des situations d'extrême précarité. Merci madame Guillemot et vous continuez avec le 596. Voilà donc le 596 par qu'on n'avait pas été vue dans le cadre du projet de loi insalubre, je le redéposera les maires font régulièrement usage de leurs pouvoirs de police pour ordonner en urgence l'évacuation des habitants d'un bâtiment en raison d'un danger pour leur santé et leur sécurité si l'extrême urgence de cette situation justifie que le maire prenne une décision rapide sur le fondement de ses pouvoirs de police et préalablement donc à l'arrêt, l'intervention d'un arrêté de police administrative spéciale, il nous paraît important de garantir aux occupants un minimum de garanties lorsqu'ils se trouvent évacuées de leurs logements, parfois sans pouvoir emporter aucune leurs affaires avec eux et on l'a vu encore malheureusement suite à de récents sinistres, il convient de rappeler en effet qu'aucun texte ne protège les occupants évacués sur le fondement des articles L 2212 2 du code général des collectivités territoriales, puisqu'il s'agit d'une urgence, il n'est pas concevable que l'autorité publique évacue des occupants de leur logement, sans qu'il n'existe aucune garantie pour eux de pouvoir bénéficier d'un hébergement ou d'un relogement, c'est pour ça que nous proposons de placer ces évacuations, je le rappelle, prises sur le fondement des dispositions dada de périls imminents du droit à un hébergement ou un relogement prévues par les articles du code de la construction de l'habitation, ça nous semble légitime. Merci madame Guillemot, monsieur le rapporteur, l'avis de commission sur ces deux amendements. Oui, madame, présente sur le premièrement je comprends difficilement la position de notre collègue Guillemot puisque je tiens à lui rappeler qu'il existe déjà une procédure d'urgence de 24 heures donc je pense que son amendement ce que nous avons évoqués lors de la commission des des lois rajoute de la complexité par rapport au au droit en vigueur s'agissant de l'amendement 596 j'en comprends la portée la pertinence, mais je me permets de demander l'avis du du gouvernement sur ce point pour nous éclairer sur les conditions d'évacuation des imams par le maire.

par ordonnance du gouvernement à revenir vers le Parlement pour régler toutes ces questions de police puisque comme vous le savez, on mélange en plus la police générale du maire avec de la police spéciale vous aviez vous-même fait référence à cette affaire-là, et donc il s'agit bien là l'accord donné demande de retrait de vos 2 heures de vos 2 amendements parce que ces hausses traiter dans le cas de l'ordonnance j'en ajouterai une remarque, en plus du sénateur Darnaud sur le 723 rectifié le pouvoir pour un maire de suspendre un bail, c'est-à-dire un contrat de droit privé, entre un propriétaire, quelle que soit la qualité du propriétaire et un locataire est quelque chose qui à mon avis et complète prince certains sur le terrain, sur le terrain juridique, en tout cas, tout ça se renvoie à l'ordonnance d'habilitation prises en cas d'élan donc demande de retrait ou, le cas échéant, même la sénatrice avis défavorable. Merci monsieur le ministre madame Guillemot pour explication de vote où nous dire si elle souhaite retirer ces amendements. Alors, bien évidemment, je ne vais pas les retirer et surtout le 1er et je voudrais dire au rapporteur, que cet amendement a été voté dans le cas de la PPL de Bruno Gilles. à l'unanimité du Sénat il y a véritablement un trou dans la raquette sur lesquels je pense vous avez pas suffisamment lu l'amendement et ici, on a tous voté. Enfin, tout ce qui était en séance, ont voté à l'unanimité des groupes PPL Bruno Jin, c'était en juin, je sais pas, ça me fait penser à à, comment il s'appelle à à des proches qui disait j'essaye de ne pas vivre en contradiction avec les idées que je ne défends pas, je ne l'impression que ça s'applique tout à fait là ce soir. Merci madame Guillemot, donc nous allons maintenant mettre aux voix, ces 2 amendements puisque madame Guillemot souhaite les maintenir, nous commençons par le 723 rectifié, donc avec un avis défavorable de la Commission et du gouvernement qui est pour. Qui est contres. On va compter, alors qui est pour.

Qui est contre. Qui s'abstient.

Voilà un article 12 c'est Madame Cukierman qui va démarrer, donc les paroles. Sur un article, merci madame la présidente, monsieur le ministre, dans quelques remarques, puisque nous allons effectivement avoir un certain nombre d'articles qui concernent le renforcement des pouvoirs de police du maire peut-être monsieur le ministre, en tout cas vous interpeller sur ce que disent. Les élus et pourrait interpellés d'abord parce que je crois, quand on parle de renforcement du pouvoir du maire un certain nombre lits voudrait d'abord puis le pouvoir existant soit effectif et court pour mener à bien ce pouvoir de police du maire déjà dans celui qui existe, il y a bien évidemment besoin d'un véritable accompagnement sur le terrain, un accompagnement en amont pour l'aide à la prise de décision bien évidemment un accompagnement au moment pour l'effectivité de, de, de, de ce pouvoir, je le disais, et puis un accompagnement par la suite pour prendre en compte les difficultés auxquelles parfois peuvent être confrontés à un certain nombre d'élus, de ne suffirait pas, en tout cas de se satisfaire par là un certain nombre d'articles telle que rédigée dans le projet de loi initial ou même tels que rots rédigé ou rajouter ici par le Sénat pour se dire que il n'y aurait plus besoin demain d'une présence de l'État qui viennent en soutien à la prise de décision des élus Loto du des élus locaux, pardon, qu'il n'y aurait plus besoin ou en tout cas moins besoin d'une présence de gendarmerie ou de police parce que à un moment donné l'effectivité de ce pouvoir de police justement et parfois mis en opposition en contradiction face à l'absence, en tout cas des personnels des forces de gendarmerie et de police sur l'ensemble de nos territoires, je crois en tout cas qu'ils ont été nombreux à l'exprimer c'est derniers mois. Donc voilà, d'une façon générale, j'ai envie dire sur cet article 10 12 pardon je voudrais décidément l'article 12 et les suivants, ce qui évitera de se répéter, ou dans les articles qui vont suivre, désolé. Merci madame Cukierman, la parole est à monsieur Olivier Jacque. Merci madame la présidente, monsieur le ministre doit faire une communication un peu particulière sur ce chapitre, dont le titre de vise à renforcer les pouvoirs de police et évoqué la problématique de la responsabilité pénale des maires lorsque officier, police judiciaire, ils exercent leur devoir, il arrive qu'en exerçant, hé bien la justice puisse se retourner contre eux, je vous donnerai à cet effet une correspondance précise d'un maire de mon département, qui sollicite le président de la République, c'est un cas récent dans mon département, dans une petite commune, le maire, rappelons-le, Jean-Claude expérimentés, très humain, vraiment très humain, pas du tout un shérif un gars violent bien un soir de 14 juillet avant le lancement du feu d'artifice, il y avait des troubles dans un groupe et donc pour l'apaiser, il y va seul et une altercation s'ensuit, il se défend, mais à 20 contre 1 en terme de témoignage, la justice a tranché cet échange de coups par un jugement de Salomon 50 50 et le condamnant à une somme substantielle de 1100 euros le maire en train de faire appel, j'en donne pas de détails, bien évidemment, le même soir, les perturbateurs sont venus à son domicile et ont ont saccagé des biens, il a porté plainte, n'ayant certainement pas assez de preuves, l'affaire a été classée sans suite, alors imaginez la désespérance de ce maire qui se retrouve dans une telle situation, bien évidemment, il a pas de police municipale, bien évidemment, il y a pas de gendarmerie sur place et la situation est pénible, monsieur le Ministre, je ne vois pas dans ce texte de dispositions qui vont permettent de prendre mieux protéger les élus qui, comme Jean-Claude prenne pleinement à coeur leur fonction. Monsieur Jacquin, la parole est à monsieur Hervé Maurey. Merci la présidente, moi je voudrais attirer l'attention du ministre sur un sujet auquel j'ai eu à connaître dans un département qu'il connaît bien et qui concerne le pouvoir de police du maire en matière d'immeubles menaçant ruine, lorsqu'il y a notamment un risque d'insolvabilité du propriétaire, vous le savez tous lorsqu'il y a un immeuble qui menace ruine le maire est tenu de mettre en oeuvre la procédure de péril qui prévoit une mise en demeure du propriétaire pour qu'il l'exécute les travaux et s'il ne le fait pas, le maire doit exécuter 2 fils ses travaux à charge de se faire rembourser par le propriétaire, le problème qui se pose, c'est lorsqu'il y a un solvabilité du du propriétaire, que celle-ci soit ou organisées et donc là on se trouve dans une situation difficile, encore une fois je, c'est un exemple qui vient du du département, dont je suis élue ou un maire n'osent pas va enclencher la procédure et n'osent pas surtout faire faire d'office des travaux sur un bâtiment, une maison, sachant très bien qu'il risque ensuite de ne pas pouvoir se faire rembourser, et donc on est dans cette situation juridique compliquée notamment et principalement pour le maire quelque part, engage sa responsabilité en ne faisant pas preuve procédé assez à travaux d'office mais qui ne veut pas le faire parce qu'il sait très bien qu'il ne sera pas remboursé et que la commune n'a pas les moyens financiers de supporter la remise en état de de cette maison, alors j'ai pas déposer d'amendement sur ce sujet, mais j'aimerais peut-être que que le ministre puisse m'éclairer sur la situation juridique et sur la et la manière dont on pourrait envisager une évolution de la législation sur ce point, peut-être dans le cadre de la navette parlementaire. Merci, cher collègue, monsieur le ministre, mes chers collègues, il est minuit presque. Et je vous propose de prolonger notre séance jusqu'à minuit et demi, afin de poursuivre l'examen de ce texte, s'il y a pas d'observation, il en est ainsi décidé. Voilà, nous poursuivons donc jusqu'à minuit et demi, alors nous passons maintenant à l'examen des amendements, le 360 tombes, ce qui n'est pas défendu le. 771 rectifié les présenté par madame Gréaume. Merci madame la présidente, monsieur le Ministre, mes chers collègues par cet amendement de suppression partielle, nous refusons que ce projet de loi sur l'aurait sûrement des élus soit vue comme une opportunité pour augmenter des amendes, ce qui est entouré ce texte vers une logique de répression qui n'est pas son but, en effet, la commission des Lois à profiter de l'examen du texte pour accroître le montant de l'amende en cas de manquement à un arrêté relatif à une fermeture d'établissement cette sanction pense, passant de 3750 euros d'amende à 10000 euros, soit bien plus du double, si nous approuvons la nécessité de donner sur certains sujets, davantage de pouvoir au maire pour faire respecter ses décisions, nous refusons que ce dernier devienne un gendarme, distribuant des amendes, nous refusons qu'il porte sur ses épaules ce poids qui pourra se retourner contre lui, par ailleurs, nous ne prenons pas que nous ne pensons pas que tout peut se régler par des amendes, ni que c'est à la hauteur de son montant que la sanction sera davantage respectés et que le trouble originel cessera l'État doit donner les moyens aux communes de faire respecter la loi, non pas par des nombreux que l'on change sur le chéquier des citoyens mais sur les effectifs et les moyens matériels que l'État assure auprès des communes en préservant et développant les services publics et sa présence où cela est nécessaire, mieux accompagner les communes, ce n'est pas augmenter les possibilités de répression. Oui, madame la présidente, il ne s'agit ici en aucun cas ne se borner à la seule augmentation des des amendes, encore moins d'exposer le maire a des responsabilités qu'il n'entendrait pas lui- même en endosser pour autant, je veux insister sur le fait que la peine d'amende prévue n'a rien de disproportionné quand on sait les conséquences pour la sécurité des personnes que peut avoir un tels comportements ou des comportements auxquels sont soumis les maires, donc bien sûr, ce sera un avis défavorable. Si monsieur le rapporteur, monsieur le Ministre, oui : avis défavorable invite défavorable. Pas d'explication de vote, explications de vote, madame Gréaume. Au parle il y a pas de répression mais n'empêche, on a quand même reçu des maires qu'ils ont été molestés. Merci, cher collègue, je mets aux voix l'amendement 771 rectifié avec un avis défavorable de la commune. Oui du gouvernement qui est pour. Qui est contres. Qui s'abstient, il n'est pas adopté l'amendement 963 et donc monsieur Darnaud va nous le présenter. teur Monsieur le Ministre. Si ces matériels c'est favorable. Elle a un avis favorable du gouvernement, je mets aux voix l'amendement 963 qui est pour.

Merci madame la présidente, madame et monsieur le rapporteur, monsieur le Ministre, la France est un beau pays, mais lorsque vous la traversée au gré des villages Oudéa mots on peut voir ça ou là des dépôts sauvages, ça peut être des frigos, des machines à laver des chauffe-eau, des voitures et Lemaire se trouve sans pouvoir de police pour pallier à ce problème et donc cet amendement vise à permettre aux maire d'utiliser leur pouvoir de police pour lutter contre ces décharges privées au même titre qu'ils peuvent le faire pour aujourd'hui des publicités qui ont marqué une pollution visuelle importante donc, cet amendement est en même temps très important pour donner le pouvoir nécessaire au maire mais pour que notre France soit encore plus belle et respecter encore plus l'environnement. Oui, et je comprends tout à fait les motivations de de notre collègue Michel Raison, pour autant il me semble que cet amendement qui vise à renforcer les pouvoirs de de police du maire pour lutter contre les décharges privées et dans l'esprit satisfait et il ne nous semble pas souhaitable d'introduire un dispositif législatif spécifique qui serait source de complexité sera une demande de retrait ou à défaut un avis d'défavorable. Merci, monsieur le rapporteur, monsieur le ministre. Oui, madame la présidente, merci monsieur le sénateur, elles ont une fois de plus, là je suis je, je, je, je vais dans le sens de ce que vous souhaitez faire néanmoins on va vers une superposition de procédure avec cet amendement dans la fatigue donc partie déjà satisfait par non seulement les dispositions telles qu'elles sont présentées par le gouvernement mais aussi par les travaux de la commission, tels que le texte a été amendé donc demande de retrait Monsieur cinéma.

envers autant le ministre-que le rapporteur Les jumeaux n'est jamais trop sûrs d'être satisfaits dans ses parce que j'ai l'habitude qu'on nous explique lorsque l'amendement convient parfaitement non non vous inquiétez pas, il est satisfait, moi je suis pas facilement satisfaits donc par principe, mais j'ai confiance en eux quand même mais je le maintiens quand même. Monsieur raison maintenant son amendement. Je propose donc de vous le de le soumettre au revoir,

Qui est contre. il n'est pas adopté après l'Arctique. Le 12 un amendement 886 rectifié, il est présenté par Madame Loisy. Merci madame la présidente, monsieur le ministre, chers collègues, cet amendement vise à donner des outils adaptés aux maires afin de mieux répondre aux risques croissants d'incendies qui sont liés, on le sait, on l'a vu malheureusement ces derniers mois aux sécheresses aux fortes chaleurs, il propose donc de donner la possibilité aux maires qui le jugerait utile d'instaurer des obligations légales de débroussaillement sur les périmètres jugés à risque de leur commune, ça concerne donc essentiellement des forêts aux abords des habitations des particuliers. Sylviana moisi, monsieur le rapporteur. Oui, madame la présidente, je ne voudrais pas abuser de la confiance de nos collègues, pas plus, notre collègue loisirs que notre collègue raison mais je puis vous assurer qu'en l'état du droit, cet amendement est est satisfait, donc ce sera une demande de retrait. Monsieur le ministre avait du gouvernement. Oui mais présentons je fais non seulement confiance et au droit et aux rapporteurs donc ma vie demande de retrait. Madame Loisier. je souhaiterais juste aucune précision parce qu'il me semblait que, actuellement, le dispositif était d'abord à la main des préfets et que c'était des périmètres qui aide étaient définies par le préfet que dans ces périmètres, effectivement, les maires pouvaient mettre en place des OMD mais s'il n'y a pas de périmètre et on le voit aujourd'hui avec un danger de risques d'incendie qui qui remonte, on a, on peut être, on peut avoir des communes un peu éparpillée qui ne justifie pas donc une une décision du préfet, donc pas de décret à l'échelle départementale ou régionale, donc est-ce que vous pouvez me répondre sur ce point, monsieur le Ministre. Monsieur le Ministre. Merci bien présente il y a pas de décret départemental, ce serait un arrêté, le cas échéant pour le, pour quel ce qu'il est possible de faire aujourd'hui bien souvent dans les faits, le maire saisissent le préfet, le préfet donne droit à ce que demandent les maires tout cas des situations, au contraire, je suis prêt à le regarder de près, ça m'intéressera beaucoup

de la police générale du maire des obligations déjà de débroussaillage sont possibles, par décision du maire en police administrative dans les faits, donc tout ça déjà satisfait. Madame Loisy vous le retirer. Merci beaucoup, donc l'amendement 886 rectifié et retiré après l'article 12 un amendement 887 rectifié madame. monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous l'avons beaucoup évoqué, les maires des petites communes rurales sont souvent isolés lorsqu'ils sont confrontés à des difficultés dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir de police, la gendarmerie a a mis en place depuis quelques mois, un dispositif de référents sécurité sur un certain nombre de territoires qui a montré beaucoup de, d'efficacité et donc cet cet amendement propose de généraliser le principe du référent sécurité qui permettrait donc aux maires de pouvoir s'appuyer sur un personnel est un professionnel qualifié qu'à même de de leçons dans des tâches de police qui ont l'a vue sont souvent de et de plus en plus délicate.

des propositions qui ont été formulées à maintes reprises par les maires consultés lors de la grande concertation et consultation du Sénat qui a donné lieu à des propositions faites par le président de la commission des lois, il y a de cela 15 jours et parmi ces ces propositions, bien sûr, l'idée d'avoir un un référent s'imposer de façon assez assez généralisé pour autant si l'idée nous paraît intéressante à creuser, elle nous paraît plus relever de bonnes pratiques locales plutôt que de faire l'objet d'une inscription dans la loi, donc si nous comprenons les motivations, si nous les partageons ce sera toutefois une demande de retrait, appelant plutôt les maires et et les autorités. de police ou de gendarmerie a engagé ces ces dispositions, donc ce sera : avis de retrait demande de retrait par Bongo : avis défavorable. Merci, monsieur le rapporteur, monsieur le ministre. merci pour cet amendement, madame la sénatrice ce matin aux invalides le général d'armée, Richard Lizurey a fait ses adieux aux armes après de longs mois et de longues années au service de notre République. Et justement, dans les grandes orientations, telles que la fameuse circulaire 100000 et pris quelques orientations sur la visibilité des gendarmes sur les capacités à retisser dans le lien armée-nation un certain nombre de choses, il y avait justement cette pratique du référent en clair une commune en face, un sous-officier de gendarmerie référent pour le maire en question et activable autant que de besoin, dans les faits c'est déjà généralisé, ce n'est pas que en Côte d'Or, que l'on connaît bien cette cette pratique, en tout cas j'espère qu'en Côte d'Or, ça fonctionne bien, le cas échéant, je me permettrai de vérifier, là aussi, le préfet de région sera ravi de puissent vérifier surtout question nous occupe beaucoup, par ailleurs, comme vous le savez, donc là-dessus, je crois qu'il est déjà satisfait, comme l'a dit le rapporteur, l'organisation des forces de sécurité intérieure ne sont pas du niveau de la loi, mais bel et bien de l'organisation décès de s'forces d'ailleurs votre amendement m'appelle cette vérification qu'il nous faudra faire autant que je crois pouvoir vous dire que ces choses sont systématiques pour les autres, gendarmerie, même s'il peut y avoir toujours quelques loupés, auquel cas on peut les on peut les corriger, il faut veiller à ce que, en zone police nationale, les choses soient aussi systématique mais, comme le disait l'sénateur Roger tout à l'heure qu'il est parti dans les zones police et souvent ensemble de, c'est le SPD qui fonctionne parce que les zones polluées sont en général beaucoup plus dense donc demande de retrait, en tout cas, vous avez eu raison de mettre un coup de projecteur sur sur cette affaire qui est, qui est quelque chose d'essentiel et qui globalement changé quand même pas mal, là les choses c'est dernières années j'en parle de manière en tant qu'ancien réserviste dans cette arme, je peux en parler longuement, mais après de longues années où les les procédures étaient très complexe dans la relation entre les élus et la gendarmerie parce que fallait systématiquement passer par les autorités hiérarchiques en clair comment groupement commandant de compagnie la les référents, mais beaucoup de bon sens, entre un gendarme ou un chef ou un adjudant on en chef est directement le maire de la commune concernée et ça pour le coup, c'est plutôt, c'est plutôt robuste et efficace, donc merci en tout cas d'avoir fait cet amendement d'appel pour nous permettent de généraliser cela, même si c'est déjà le cas de veiller à ce que soit bien faire zone police.

par les uns comme par les eaux, donc je pense qu'on a là un bel outil qui pourrait répondre à beaucoup de difficultés sur nos territoires, merci donc. Merci, cher collègue, l'amendement 887 rectifié et retiré nous passons à l'article 13 d'abord, l'amendement 361 qui n'est pas défendu le. 91 rectifié, il est présenté par Nathalie Delattre. Chers collègues, merci madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues en 1er vu mieux vous dire qu'en qu'en Gironde cet art qui n'est pas vraiment voulu par une majorité des mères qui pense que, en la matière, il était plutôt utile d'avoir le préfet comme filtre cependant cet amendement exploite le sujet en s'intéressant à un autre volet qui est l'ouverture de ces établissements de saisie débits de boisson, sur lequel le maire n'a même pas le droit aujourd'hui d'émettre un avis consultatif, alors que lors de la déclaration, le maire est en charge de récolter les différents justificatifs et de vérifier que le dossier complet, une fois que ce dossier complet, le maire doit délivrer le récépissé à la personne qui souhaite rouvrir cet établissement dans les 3 jours, il doit transmettre au procureur de la République et au préfet du département copie intégrale de la déclaration et c'est tout, pourtant, lors de ce transfert le pourrait avoir le droit de formaliser un avis consultatif sur le dossier et mettre ainsi en cohérence les pouvoirs qui lui sont donnés dans cette dans concernant la fermeture des établissements avec un avis sur l'ouverture de préciser que dans le cadre d'une demande de transfert d'un débit de boisson d'une commune à une autre, le préfet a d'ores et déjà l'obligation de consulter le maire de la commune où le débit de boissons va être installée, mais comme le propose aussi cet amendement leur avis ne lie pas le préfet il vous l'aurez compris dans un souci de cohérence, il est proposé que le maire puisse donner un avis sur une implantation débits de boisson, de 3ème et de 4ème, catégorie et des établissements pourvu de la petite licence restaurant ou de la licence restaurant, décision qui impacte parfois lourdement la le territoire de ça quoi. Merci, merci madame De Lattre, monsieur le rapporteur, avis de la commission. Oui, madame la présidente, je voudrais juste rappeler à notre collègue Nathalie Delattre, même si je comprends encore une fois, les raisons de de cet amendement que l'ouverture d'un débit de boisson et soumise à un régime de déclaration administrative et non d'autorisations administratives, en conséquence, le refus d'ouverture d'un débit de boissons ne s'apprécient pas en opportunité, le préfet une compétence liée et se contente de vérifier la régularité et la situation du déclarant que le respect de la législation applicable aux débits de boissons, en particulier des quotas d'installation sur le territoire de la commune, dans ce contexte, l'avis du maire n'a, n'aurait aucune valeur ajoutée, pardon, notons en outre qu'un avis simple qui ne lirait pas le préfet ne serait pas de nature à renforcer les pouvoirs de police du maire, ce sera donc un avis défavorable. le rapporteur, monsieur le ministre. Oui, madame la présidente, même avis que que le rapporteur, j'ajouterai que même peut-être Madame la cette risotto qu'en partie, il peut être satisfait si l'on regarde que parfois ce lieu sera un ERP un établissement recevant du public, elle a, par ailleurs, vous avez les procédures que vous connaissez sur sur les ERP donc demande de retrait ou avis défavorable. Vous maintenez l'amendement donc l'amendement étant maintenu, je le mets aux voix donc il un avis défavorable de la Commission et du gouvernement qui pour. Qui est contre. Qui s'abstient, il n'est pas adopté, nous avons 5 amendements faisant l'objet d'une discussion commune le 1er de 489 rectifié bis est présenté par Monsieur Merci madame la présidente, monsieur le ministre, chers collègues, avec plusieurs collègues, nous nous sommes interroges effectivement sur cette disposition qui tendrait à confier au maire, la police spéciale des débits de boissons, une compétence pour pouvoir enregistrer les déclarations des mi-boissons et puis pour aussi pouvoir octroyer des autorisations plus tardif pour jusqu'à un certain horaire mais quel est véritablement l'intérêt de le doter d'une compétence lui présentera la matière les problèmes de police sur les débits de boisson requiert la présence des forces de l'ordre que ce soit la gendarmerie en zone rurale, la police en zone urbaine et à qui ces organes vont en référer, bien entendu, au préfet, puisqu'ils sont sous l'autorité du préfet ne sont pas sous l'autorité du maire et donc il convient que ce soit le préfet qui l'assure d'autant plus que on voit bien qu'il y a quand même dans ces dispositions, la nécessité d'une approche qui soit globale et cette approche globale, seul le préfet peut l'exercer, puisqu'il a une vue globale sur l'ensemble du département et non pas simplement une vue partielle au cas par cas et si l'on veut véritablement qu'il de l'équité dans le traitement, sur un même département vis-à-vis de situations d'incivilité ou de difficultés, hé bien c'est vraiment le préfet qui a la possibilité de l'assumer, donc c'est le sens de cet amendement qui vise à supprimer 11 alinéa 2 de cet article pour faire en short que hé bien le le dispositif actuel puisse perdurer. monsieur Calvet, la parole est maintenant à monsieur Cabanel pour défendre le 212 rectifié. Merci madame la présidente, monsieur le ministre, chers collègues, il est proposé par cet amendement de remplacer le délai de fermeture de 2 mois maximum par un délai de 2 mois reconductible afin de permettre au préfet, au maire de reconduire le délai de fermeture si aucune solution n'a été trouvé pour mettre fin au trou pour l'autre à l'ordre public, provoquée par le débit de boissons, car il arrive bien souvent que la fermeture de 2 mois ne suffisait pas à faire rentrer dans l'ordre des comportements illicites. Si Monsieur Cabanel, Madame Lavarde va défendre le 118 rectifié bis. Et le 119 en même temps, puisque pour ces 2 amendements, je suis le porte-parole de notre collègue Philippe Dallier, qui les a déposés, donc en l'état actuel du texte, l'article 13 du projet de loi vise à transférer un des pouvoirs du préfet visées à l'article L. 33 32 15 du code de la santé publique 1000 transferts uniquement le petit 2, à savoir la fermeture administrative pour trouvera là on voudrait public l'amendement 118 lui vise aussi à transférer au maire le pouvoir prévues au petit I du même article du code de la santé publique, à savoir la fermeture administrative en cas de non respect des lois et des règlements et l'amendement 119 étaient en fait un amendement de repli, puisqu'il vise à restreindre le Champ d'application de ce petit hein uniquement aurait au non respect des règlements municipaux. Merci Madame Lavarde enfin, le 772 rectifié, il est présenté par Monsieur Gay. Merci madame la présidente, monsieur le Ministre, mes chers collègues, bon on aura débat sur David de Poisson donnera notre avis sur les quatre amendements avant, nous nous posons une question, c'est : jusqu'où va s'arrêter la liste à privé. On pense qu'il faut supprimer les alinéas sur la question de la musique parce que on va, on va voir, il faut rentrer dans le dur, c'est quels moyens après on donne au maire pour faire respecter tout ça. C'est une question. Parce que je partage la philosophie de notre collègue Michel Canevet qui a défendu le le 1er rendement sur le débit de boissons, comment faire après pour faire respecter. Ce nouveau pouvoir du maire. Si on n'y met pas les moyens. Avec la présidente assassine ou et donc nous sommes élus en Seine-Saint-Denis. Il y a des questions autour des débits de boissons, mais on peut donner le pouvoir aux maire. Oui, les forces de l'or pour l'accompagner pour faire respecter la loi. Je vous pose la question Monsieur le Ministre, va voir la police de sécurité du quotidien. à part aux informations à la télé, on les a pas vu nous, sur le terrain et les élus municipaux et locaux non plus non, mais je dis ça parce que quand on est habitant par exemple en Seine-Saint-Denis. On a moins d'officier de police du judiciaire qu'à Paris, moins aux policiers tout court qu'à Paris et après, si en plus vous arrivez à aller jusqu'à la mort, après qu'il soit condamné, il faut qu'il passe au tribunal, il y a moins de juges que partout ailleurs. Donc je dis ça parce que on il faut pas qu'on ait un débat hors sol Alors on peut avoir le débat sur débits de boissons, on peut la voir et on n'est pas fermée sur cette question, on va donner notre avis après après évidemment, monsieur le rapporteur, Monsieur le Ministre, mais franchement, ajouter la question de la musique là-dessus, ça nous paraît inopportun, donc nous proposons vraiment de supprimer ces deux alinéas je vous remercie. Merci, cher collègue, alors nous passons maintenant à l'avis de la commission, monsieur le rapporteur. Oui, madame la présidente, s'agissant de l'amendement présenté et défendu par notre collègue, collègue, je ne vais pas revenir sur les arguments que j'ai déjà évoqué lors du précédent amendement, donc ce sera un avis défavorable, s'agissant de l'art, l'amendement pardon 212 de notre collègue Cabanel, je voudrais rappeler que la loi prévoit 3 motifs de fermetures de débits de boissons et il serait donc peu cohérent de prévoir une possibilité de prorogation que pour l'une d'entre 2, s'agissant des amendements 118 et 119 de notre collègue Philippe Dallier, l'amendement 118 qui vise à donner la possibilité aux maires de fermer des débits de boissons, non seulement pour des motifs d'ordre public, mais également en cas de non respect de la réglementation en vigueur, en vigueur, ce sera un avis favorable en revanche un avis défavorable au 119 enfin sur l'article 772 j'entends complètement les arguments avancés par notre collègue Fabien Gay, à ceci près que c'est un débat qu'on va pouvoir avoir tout au long. De ces discussions autour des amendements sur le pouvoir de police des mers, puisque c'est une faculté et malheureusement ne trancheront pas nécessairement la question des moyens de de sécurité donc il s'agit de mettre en cohérence, ce que nous avons appelé de nos voeux sur les pouvoirs de police des mers et ce sera donc un avis défavorable. Merci, monsieur le rapporteur, monsieur le ministre à vie du gouvernement. Oui, madame la présidente, ils ont fait l'objet d'une discussion commune mais, enfin, mine de rien, ils ne disent pas tout à fait tous la même chose, un court instant pour bien s'assurer qu'on disent tous la même chose : 489 rectifié votre un moment même la présidente défendu par par votre collègue, je rappelle juste qu'au final, il est déjà satisfait dans la mesure où je vous regarde en même temps, dans la mesure où cette faculté qui est ouverte au maire n'est qu'une faculté. Le maire demande aux préfets de se voir attribuer ce pouvoir de police administrative ou pas, donc, dès lors que c'est une liberté, je pense que le maire qui a envie de le faire, le fait est le maire qui n'a pas envie de le faire et le fait pas, ça me semble la meilleure des choses et la meilleure des garanties que l'on puisse faire, mais vous avez raison, il faut le rappeler parce que sinon ça mais le maire potentiellement dans une seringue et ça c'est pas une bonne chose. Donc là on garde ce principe de liberté et en plus, comme vous le savez, tout cela est conditionné dans le temps, parce que là on est sur des choses, on l'a peut-être un peu, dit-on, DG enfin avec la commission des lois, en commun avec le gouvernement, on assume aussi d'aller sur le terrain d'une forme d'expérimentation parce que souvent on a renforcé le pouvoir de police des mers, on a rarement fait descendre de la police administrative du niveau du préfet, au maire et dans la protection de la proximité, l'ère engagement et proximité, l'un dans le mot proximité c'est pas que de la décentralisation, la proximité, c'est aussi la déconcentration de pouvoir du corps préfectoral vers le maire en tant qu'agent de l'État, donc là on a, à mon avis quelque chose qui, qui est déjà satisfait mais s'était utile, à mon avis, que de rappeler sur le 212 rectifié de monsieur Cabanel ah oui, alors si c'est intéressant, il faut garder quand même la capacité de rouvrir, je m'explique : vous prenez un arrêté pour fermer pendant 2 mois. Syrie enfin et vous ne pouvez pas reprendre un arrêté pour faire 4 mois

pour le coup, là en terme d'excès de pouvoir et de fragilité de l'acte, on serait évidemment complètement dedans, mais rassurez-vous, c'est pas de moi, et puis ensuite c'est fini, c'est 2 mois et puis si on constate encore mais faut refaire le constat mais c'est ce qui protège aussi la la la démarche du maire, comme l'amendement précédent. Madame la présidente demande de retrait si vous êtes d'accord, mais la précision était à mon avis là aussi importante sur le 118 rectifié bis monsieur le rapporteur, vous avez bien lui favorable dansez sur suivant 68, vous avez mis un avis favorable alors je, je, mais 20 heureusement je mettrais un avis défavorable, parce que l'enfer est pavé de bonnes intentions, typiquement sur cet amendement, je ne fais pas un cas mais je pense qu'il faut quand même qu'on fasse attention à protéger, nous nous nos la frontière entre police administrative et police judiciaire est une frontière ténue je le 1er au sénateur Dallier au président d'alliés de regarder de près, son amendement est en déplacement, c'est pour ça qu'il ne peut pas présenter ce soir est bien sûr excusez, je lui en un retour, c'est compliqué de demander à un maire de commencer à contrôler. D'autres critères que l'ordre public, droit du travail. L'hygiène. la consommation de stupéfiants dans un débit de boisson ou un lieu de restauration, vous voyez, là, on passe d'un schéma de police administrative, on regarde la question de l'ordre public. Et uniquement de l'ordre public comme un membre du corps préfectoral, le ferait et donc le juge administratif bien sûr référé-liberté référé pourquoi avec, c'est de pouvoir enfin tout ce que vous connaissez est efficient. Mais si vous commencez à aller chercher d'autres bases légales pour justifier une fermeture, c'est plus de l'administratif. c'est un début de constat judiciaire, bon et là pour le coup, on revient avec le maire en tant que OPJ mais comme vous le savez l'OPJ ne peut pas et constaté et en même temps condamné. Sauf pour les contraventions, code de la route etc bon, donc là je pense qu'on s'achemine dans quelque chose que je que je vois bien pour des raisons éminemment locale pour lequel elles ont pu être proposées mais demande de retrait parce que je pense que là, on ne fait pas que des choses utiles et facile pour les élus et avec une fragilité à mon avis qui sera vite qui sera vite démontré à la première 1er contentieux venu une fois plus mélangés police administrative et police judiciaire dans nos dans nos débats et dans nos amendements et dans nos votes dans vos votes et moi dans mes avis à mon avis n'est pas n'est pas une bonne chose, donc : demande de retrait sur le 119 rectifié. Pour le coup, là, monsieur le rapporteur, vous avez émis un avis également favorable, si j'ai bien tout noté favorable, défavorable, défavorable, bon alors là je suis honnête avec vous, je ne comprends pas, on rajoute la la l'inspiration sur l'arrêté municipal. Pour le.

moi je donc plutôt avis défavorable, pardonnez-moi mais je, je, je ne comprends pas complètement l'opportunité mais c'est certainement la fatigue avec cette heure avancée, monsieur le sénateur sur vos 2 remarques bon sur la musique, ce n'est pas le gouvernement qu'il n'introduit, c'est la commission, on y reviendra dans les débats là-dessus sagesse mais je vois bien les conditions est. Ce n'est pas le gouvernement qui a introduit. Moi j'ai pas dit ça, je dis juste que je, je, j'ai ma paternité et le président à la sienne et donc la Commission répondra et réexpliquant j'imagine ce pourquoi la question de la musique est intervenu dans les débats, moi je le sais mais c'est pas à moi de rapporter les travaux de la commission par définition sur les moyens pour appliquer je vois votre interpellation. Si j'en reste à l'amendement, enfin surtout à à l'article 13 l'intérêt l'de de la police administrative, c'est qu'elle est souple pour le maire et que c'est une décision et qu'une décision, c'est un arrêté non mais dans les. J'étais maire, je vois bien comment ça fonctionne, donc la réalité, c'est que ce sont des décisions qui sont d'une décision, une très grande souplesse et si vous avez un débit qui débute Bresson, par exemple, qui décide de rester ouvert malgré l'arrêté là c'est pas le maire qui engagent l'action publique, hein, c'est le parquet, lorsque vous avez un arrêté de police administrative qui soit préfectorales ou qu'ils soient municipales s'il n'est pas appliquée, on retombe dans ce que vous connaissez par ailleurs en tant que législateur sur l'application du droit et donc, par définition, ben c'est l'action publique qui se déclenche, c'est le recours à la force publique, le cas échéant, c'est éventuellement des articles 40 qui peuvent être déclenchées, je veux dire, ça j'ai j'ai tenu à cette ligne-là et d'ailleurs la présidente Assassi. un peu partout, les effectifs sont en tension parce que vous n'êtes pas sans savoir, mesdames, messieurs les sénateurs, que les policiers, les gendarmes accomplissent aussi des missions nouvelles sur le terrorisme sur Lens du public, on l'a bien vu, donc non, non, mais c'est plus j'ai porté l'uniforme, non je ne méconnais pas la difficulté dans ces unités non non j'ai pas tout fait, mais je, je, je témoigne parce que je pense que c'est bien aussi de le faire, je dis juste, c'est je vois bien votre débat sur les moyens, ce que je dis, c'est que ça, ce sont des moyens concrets, juridiques qui permettent d'avancer. Merci monsieur le ministre, je vous propose maintenant de procéder au vote sur ces amendements. Je veux dire. Alors avant, il y a toute une série d'explications de vote, nous allons commencer par Monsieur Durand. Merci madame la présidente, écoutez je profiterai de de ce premier amendement mais ça aurait pu intervenir sur d'autres pour un propos un peu général sur sur les pouvoirs de police pour avoir rencontré les, les, les élus et leur avoir soumis le texte ces articles et c'est et ses intentions, ce que demandent les élus locaux s'agissant des pouvoirs de police, c'est moins d'en avoir plus que de pouvoir déjà correctement faire parce qu'ils ont à faire la question de l'effectivité de leur pouvoir de police et centrale, c'est derrière la question du lien avec la gendarmerie avec la police, avec le procureur, la capacité à articuler intelligemment toute cette chaîne derrière la décision prise par les local et donc ce que nous disons à l'étude de ces, de ces amendements et cet article et ces articles c'est : faut-il vraiment donner de nouveaux pouvoirs s'il n'y a pas de nouveaux moyens et faut-il vraiment généré désespoir en matière de pouvoir de police, si on n'est pas en capacité de sécuriser la capacité pour les maires d'aller au bout des intentions qu'il manifeste en matière de pouvoir de police, faute de quoi, c'est un peu le miroir aux Alouettes, faute de quoi, on peut un peu tromper son monde, faute de quoi, on peut même mettre une pression inutile sur des maires sur lesquels on va faire peser de nouvelles responsabilités alors qu'il peine déjà assumer celle qui leur incombe aujourd'hui. Merci Monsieur Durand dans la série de demandes d'explication de vote j'ai Monsieur Gay. Merci madame la présidente, nous je partage en l'intervention de notre collègue du Rhin, je le dis à monsieur le rapporteur a Monsieur le Ministre. On a sincèrement cette réponse, vous avez raison, mais c'est pas le moment de parler des moyens oui mais je je reprends prenant des cas très pratique. Demain, si vous offrez cette possibilité au maire la population va se tourner vers le maire, et donc il va prendre un arrêté mais il n'aura aucun moyen de l'appliquer et on va créer des disparités parce qu'il y aura des villes qui auront les moyens parce que seront par exemple une police municipale importante et puis à côté, une ville qui n'aura pas les moyens, mais qui, pas de police municipale, mais qui y compris cherche les effectifs et je redis, bon, désolé, on a ce tropisme mais dans le 93 on a déjà pas assez de moyens dans la police pour assurer les missions régaliennes, alors qu'on sait sur la fermeture des débits de boissons et qui est une réalité, par exemple, qui peuvent être des nuisances très fort pour les populations. Plusieurs jours par semaine, donc on va créer de l'espoir et en fit au final on ne réglera rien et ce sont les élus locaux qui vont se retrouver face à cette situation, donc franchement. On votera donc l'amendement présenté par Madame l'État et ses collègues puis évidemment le note sur la suppression de ces alinéas qui n'apporte en vérité qu'une vraie fausse

à monsieur Calvet nous passons maintenant au 489 rectifié bis vous le retirer, je vous remercie le 212 donc ce monsieur Cabanel est retiré. Le 118 rectifié bis Madame Lavarde. Alors je vais maintenir le 118 rectifié bis et je vais retirer du fin notamment, parce qu'on va être le 119 visait à dire que si jamais on considérait que le maire n'était pas en capacité de pouvoir juger de l'ensemble des lois et règlements donc ce que j'ai bien compris dans votre exposé, Monsieur le Ministre on l'y autoriser quand même enfin lui donner la capacité de pouvoir gérer les arrêtés municipaux qui est de son pouvoir, puisqu'il les a écrits et entre guillemets, fait voter par son conseil municipal, donc c'était l'objet de la 219 est peut-être mal écrit, donc on peut peut-être laisser le 118 dans la navette et comme ça vous pourrez reprend l'idée du 119 c'était ça qui posait problème ou voilà donc je laisse le 118 qui l'arsenal est favorable de la commission. Alors merci madame donc je mets aux voix l'amendement 118 rectifié ce qu'il y a donc un avis favorable de la commission et une demande de retrait du gouvernement qui est pour. Qui contres. Qui s'abstient l'amendement est adopté, donc le suivant est retiré et le 772 rectifié je procède au vote sur cet amendement, qui a un avis défavorable de la commission, mais une sagesse du gouvernement qui est pour. Qui est contres. qui s'abstient, il n'est pas adopté, il reste. 2 amendements, avant de conclure : peut-être on termine cette partie. Vous êtes d'accord. Allez, on continue, on va vite monsieur le roi pour le 576 rectifié bis. Je vais aller très vite, madame la présidente, ministre, mes chers collègues, ben écoutez, ça rentre dans le même état 10 prix l'objet de mon amendement et d'autoriser le maire à réglementer les ouvertures de commerces, de nuit, lorsque le fonctionnement ces établissements compromet le bon ordre et la tranquillité, la tranquillité Merci, cher collègue, avis de la commission. la vente d'alcool à emporter sur certaines zones entre 22 heures et 8 heures du matin, ce qui vise, entre autres, les épiceries de nuit, donc c'est une demande de retrait ou à défaut un avis défavorable. Si Monsieur le Ministre, mais ma vie mais ma avis même présidente, monsieur le sénateur vous le retirer. Il est retiré, le 880 94 rectifié Yves. Présenté par Monsieur chaise. La présidente, monsieur le ministre, l'amendement que je présente, vise à permettre à la police municipale d'intervenir sur demande des propriétaires ou des exploitants de terrains dès lors que ces derniers s'occupé par des personnes qui ne respectent pas les principes d'accès, de libre circulation des personnes autorisées de sécurité de sûreté et de tranquillité des lieux actuellement le code de la sécurité intérieure permet de faire appel à la police municipale pour les squats dans des immeubles d'un d'habitations, l'objet de l'amendement et de l'étendre au terrain donc d'exploitation. Oui. Cet amendement en quittant autoriser les agents de police municipale a procédé à l'évacuation d'office d'un terrain privé sur simple demande du propriétaire, si on peut comprendre l'objet, il est évident que cette disposition aurait principalement vocation à être appliqué dans la pratique à l'encontre des occupations illicites des gens du voyage, comprendre, encore une fois la la portée, toutefois, à moins qu'elle n'ait été autorisée par un juge l'évacuation d'une occupation illicite d'un terrain public comme privé constitue une mesure de police administrative et doit à ce titre être entouré d'un certain nombre de garanties destinées à en assurer la proportionnalité, c'est ainsi que l'évacuation d'office des campements illicites ne peut être mise en 9 qu'à l'issue d'une procédure encadré par le législateur, après mise en demeure par le préfet et garantissant le droit au recours effectif enfin au-delà de ces difficultés juridiques que nous n'avons pas jugé souhaitable de confier aux seuls agents de police municipale sans appui de la police ou la gendarmerie, le soin de procéder à des évacuations d'office, il ne serait pas à notre sens opportun de permettre à ses agents, qui ne sont pardon ni formés, ni équipés à cet effet de procéder seul à ce type de mesures coercitives, ce sera donc un avis défavorable. Merci, monsieur le rapporteur, mais ma vie même avis mais la présidence à l'heure, le monsieur boeuf cher demande la parole. La là-dessus. La présidente, monsieur le Ministre, c'est quand même un vrai sujet, moi j'entends bien que la police municipale pour déloger les gens du voyage, c'est sans doute pas la bonne solution, on va en convenir pour la sécurité de tous, simplement il y a là un vrai sujet et vous pouvez pas l'ignorer, donc moi ce que j'aimerais, monsieur le Ministre, si vous prenez l'engagement, à défaut, que ce soit traité ici dans cet hémicycle que vous preniez le temps de gérer le sujet à l'Assemblée nationale. Merci Monsieur HR Madame Schillinger demandé la parole. 200 jeunes sur un terrain privé, où la police n'a pas pu évacuer et juste, il y avait enfin communes impactées, la musique était tellement forte, il se mettait même eux-mêmes en danger, donc à un moment donné, il faudra trouver des solutions pour aussi sécuriser les jeunes qui vont sur des terrains privés mais voilà c'est c'est parmi d'autres sujets. Merci, cher collègue. Je vais maintenant mettre aux voix, cet amendement, s'il n'y a plus de demandes d'explications de vote avec un avis défavorable de la commission.

on a la difficulté de trouver le propriétaire, lui-même, le propriétaire ne peut pas faire la démarche, et il faut que le maire puisse se substituer à l'ensemble des propriétaires pour maintenir l'ordre, donc je retire mais avec une demande vraiment d'Express, de revenir sur ce sujet très rapidement. Merci monsieur chaise, cet amendement est donc retiré je mets aux voix, l'article 13 qui est pour. Qui compte. Qui s'abstient, il est adopté, mes chers collègues par courrier en date de ce jour Monsieur Bruno Retailleau, président du groupe, les républicains demande de retrait de l'ordre du jour du mardi 22 octobre après-midi de la proposition de loi tendant à réduire le nombre de sièges à pourvoir au sein des conseils municipaux des communes de moins de 500 habitants en raison d'un nombre insuffisant de sièges pourvus à la suite d'un 2ème tour de scrutin municipal acte et donné de cette demande, je n'ai été saisi d'aucune observation sur les conclusions de la conférence des présidents, elles sont donc adopté mais, chers collègues, je vais lever la séance, nous avons examiné 102 amendements au cours de la journée, il reste 320 et 327 amendements à examiner sur ce texte prochaine séance, mercredi 16 octobre à 15 heures pour les questions d'actualité au gouvernement, la séance est levée.